La séance est reprise. Et appelle l'examen des articles non rattachés du projet de loi de finances pour 2023, tous les crédits indicateurs de performance afférents mission été examiné le Sénat va désormais statuer au sein de la seconde partie du projet de loi de finances sur les articles qui porterait capitulation de ces crédits indicateurs. Je vais donc appelé les articles 27 à 31 et les États B A. Et j'ai qui leur sont annexés. La direction de la séance à procéder à la rectification des États annexée de manière à tenir compte des votes intervenus lors de l'examen de la seconde partie du projet de loi de finances je mets donc d'abord on voit l'ensemble le consul, l'article 27 de l'État qui est annexée qui est pour.--

Alors concernant cet article 32. Qui fixent les plafonds des autorisations d'employes de l'État pour 2023, en rappelant que précédemment. L'ensemble des missions. Des Des 33 mission qui ont été étudiées. Précédemment pour la deuxième partie. Les crédits au total s'élève à 500, à plus de 567 milliards d'euros

Plus de 272.000. Économie, Finances Souveraineté industrielle et numérique. Plus de 125.855 emplois avec une baisse néanmoins de moins 444. ETPT et aussi la justice. Plus de 92.000 emplois, c'est je cite les principaux. Sans oublier que les articles suivants. 33. Aussi les plafonds des employes des opérateurs de de l'État. plus de 406.000. Emplois. Notamment avec la mission recherche enseignement supérieur de l'or, de 256.000 emplois. Donc je soutiendrai. Cet article, merci. Merci monsieur Savoldelli.-- Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Nos collègues Marc midi a beaucoup parlé d'emploi.-- Mais je ne sais pas si libre du bon côté.-- Parce que si j'ai bien compris. Ce projet de loi de finances 2023 devaient avoir le mérite pour la droite sénatoriale. De traduire en actes un amendement. Mes chers collègues, que vous avez adopté lors de la loi de programmation pour 2023 2027.-- Dans cet amendement vous visiez à réduire. Donc la droite au sénat de 5 pour % les agents de l'État. Un amendement qui sabrer oh allez 120.000 postes de fonctionnaires d'ici 2027.-- Donc une trajectoire de réduction de l'emploi public jamais réalisé jamais tenues et d'une brutalité sans précédant. Aucune réduction là aucune réduction Arctique 32 Arctique 33 les aucune réduction dans le poids n'a été proposé concernant l'état ni par la commission ni par l'auteur des amendements question ni par ceux qui l'ont voté. Hé ben oui vous faites un constat, personne n'a trouvé de postes superflus. Dans le cadre de ce budget qui prévoit quand même près de 19.000 équivalents temps travaillé supplémentaire par rapport au budget précédent. Je dis ça parce que pour les opérateurs de l'État. Les amendements proposés qui vont être débattus ici et et. Par enfin et délibérée par notre hémicycle et de majorer les employes du Conservatoire du littoral. Allez, nous on va aller voter. De l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, on va aller voter pour l'agence publique pour l'immobilier de la justice, on va aller voter et on va voter aussi les employes de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions. Franchement.-- Enfin je ne sais pas comment vous vivez ça, vous êtes peut être bien dans votre peau mais on ne peut pas avoir décidé de vouloir supprimer 120.000 emplois. Et puis après dans des amendements rajouter des emplois, des emplois des emplois.-- Il y a un moment il y a une petite contradiction qui doit pas être facile à digérer.-- Merci Monsieur le Ministre, vous avez un amendement cet article 32.-- qui ont un impact sur le plafond des autorisations d'employes de l'État pour 2023. Si je dois résumer les principaux mouvements le plafond d'emplois du ministère de la justice augmente de 691 qui va en temps plein. C'est en fait le choix qui a été fait de renouveler pour 3 ans, des contrats qui avait été fait pour trois ans, notamment sur le volet justice de proximité et lutte contre les violences intrafamiliales ces contrats arrivés à échéance au mois de juin dernier il a été décidé en juin dernier de les renouveler pour 3 ans. Il fallait pour cela attendre que le PLFR. Que nous avons adopté, relève le plafond d'emplois pour faire la coordination en PLF on ne pouvait pas le mettre en PLF tant que le PLFR n'avaient pas voté ces contrats supplémentaires. Pour la lutte contre les violences intrafamiliales et la justice de proximité. principal mouvement qui est celui du ministère de la justice. Ensuite il y a pour ce qui est du ministère de la transition écologique des effectifs à la fois qui diminue mais qui sont les effectifs qui font suite au transfert vers les régions, la gestion des sites Natura 2000 et de la gestion des routes et des personnels de la collectivité européenne d'Alsace et de l'Eurométropole de Strasbourg il y a aussi des plus au ministère de l'Écologie. On rajoute notamment 5 postes à la creux. La Commission de régulation de l'énergie dont on imagine bien et vous imaginez bien, en ce moment qu'elle est particulièrement mobilisée particulièrement sollicités. Vu les les la crise que nous connaissons aujourd'hui sur les prix de l'énergie si postes également pour renforcer les cross sur la surveillance et le sauvetage en mer et puis enfin il y a des redéploiements au sein des administrations territoriales de l'État. Donc il sait que c'est c'est Qui méritent moins d'être détaillé.-- Merci, monsieur le Ministre, quel est l'avis de la commission. Monsieur le rapporteur général sur cet amendement du gouvernement. Voilà. La commission n'a pas d'avis mais le rapporteur général un avis je dis dit n'a pas d'avis parce que. Nous n'avons pas eu à nous prononcer sur. Cet amendement, comme l'a dit le ministre. Néanmoins il tire les conséquences d'un certain nombre de décisions qui ont été prises. le l'exercice 2022 et. Pour je ne sais pas si ça rassurera mais pour rassurer. Néanmoins, notre collègue Pascal Savoldelli, c'est effectivement un certain nombre de créations de postes d'ajustement et de redéploiement et il faut également que chacun assume sa cohérence sur des dispositifs qui. Parfois, ou des votes qui entraîné des créations d'emplois. On n'est pas là pour revenir sur des votes qui sont acquis. Donc, à titre personnel un avis de sagesse.-- Oui pour. Explications de vote. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, oui je je je vois dans la liste des postes effectivement aussi des situations conjoncturelles pour répondre à notre collègue ça le Je pense notamment à ce qui concerne le cross mon est mer du Nord. Vous le savez, il y a énormément de traverser en ce moment et le cross qui fait la surveillance de cet espace dans le Detroit a besoin d'emplois. C'est d'ailleurs été l'objet d'un amendement que nous avions déposé avec Christine Lavarde mais qui a été reconnu, article 40, en échange bien sûr en discussion avec le ministère sur cette question, donc je vous remercie monsieur le ministre d'avoir pu intégrer. Ces 6 emplois. je vais, je vais donc mettre aux voix cet amendement. Mais Savoldelli pardon.-- Oui merci madame la présidente, monsieur le ministre.-- Bah, Monsieur le Ministre, ça commence bien parce que nous on va voter pour votre amendement. Parce que là franchement.-- J'ai écouté mon ont collé grappin mais on on n'est pas sur les mêmes échelle là ou quoi. Vous avez fait voter 120.000 emplois de moins.

Mais en gros on en supprime 120.000 il y a quelques jours là on va chipoter sur des justement qui sont quand même se solde au positif. Vous me direz si je me trompe.-- Et puis de l'autre côté vous avez enfin de l'amendement pour ajouter des emplois publics. Enfin enfin franchement. Franchement. Faudrait que ça considère les les citoyens les citoyennes ça.-- C'est une belle image de la politique.-- Mais en tout cas moi j'en doute. S'il n'y a pas de madame Lavarde. merci madame la présidente, je voudrais saisir l'occasion qu'on ajoute les cinq ETP. Pour la Commission de régulation de l'énergie, qui ont été évoqués mercredi. pour dire que, à l'occasion du débat que nous avons eu dans cet hémicycle sur l'article 42 terre. La ministre a pris l'engagement de nous fournir chaque mois l'état des subventions versées par les fournisseurs aux consommateurs, mais il y a certaines des données qui nous intéresse aussi qui ne sont pas dans le giron de la Commission de régulation. C'est notamment le niveau de la contribution la contribution de la rente infra-marginal. J'ai compris que ça c'était suivi par un autre ministère que la transition donc nous aimerions aussi ajouté ces données et comme je pense qu'elles viennent de chez vous. La demande est faite. Très bien, s'il n'y a plus d'autre explication. Comme votre vais mettre aux voix cet amendement du gouvernement avec un avis favorable du rapporteur qui est pour.-- Qui contrôle qui s'abstient il est adopté. Je me vois l'article 32 qui est pour. Qui est contre qui s'abstient adoptée à l'article 33. Nous avons trois amendements identiques et on commence par. Qui Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, je présente. Un amendement à l'initiative de notre collègue Jean-Claude Tissot qui vise à renforcer les effectifs de l'Agence Bio. En effet il y a on constate actuellement une perte de vitesse dans le développement du bio qui est pourtant au coeur de la feuille de route du gouvernement de beaucoup d'élus sur ces bancs, si nous avons augmenté le Fonds Avenir Bio prévues par ce projet de loi de finances. Nous avons également à mettre en oeuvre la loi Egalim à augmenter l'offre bio dans les cantines il nous semble donc indispensable d'augmenter le budget alloué aux ressources humaines de l'Agence Bio, cet amendement propose donc de rehausser de 20 ETP le plafond des employes de l'Agence Bio pour pouvoir couvrir l'augmentation des dossiers à instruire dans le cadre du fonds de structuration Avenir Bio et de mettre en oeuvre efficacement les actions de communication et de soutien au développement territorial de l'agriculture biologique, cet amendement prévoit donc d'une un relèvement du plafond d'emplois des opérateurs du programme 149 de 20 ETP pour les fléché vers l'Agence Bio en espérant que si cet amendement être adopté. Le gage sera levé par le gouvernement, car le but n'est pas de baisser le plafond d'emplois sur le programme de 106 qui constituent le gage de cet amendement, je vous remercie.

L'organisme de la l'Agence Bio reste sous-financé se trouve en difficulté pour mener véritablement à bien sa mission et nous sommes dans un contexte de plus en plus d'agriculture adopte le mode de production bio, même si on sait que c'est une une agriculture qui aujourd'hui et tenter difficulté c'est à la fois une bonne Buffel puisque ce mode de production porteur de sens permet de respecter l'environnement. Le bien-être animal la santé des consommateurs et de ne pas s'exposer à des pesticides. Néanmoins, on constate un ralentissement de la demande, ce qui crée un déséquilibre et les difficultés économiques pour les producteurs alors que les filières conventionnelles lorsqu'elle rencontre ce type de difficultés conjoncturelles, se voit aidée par différents mécanismes, publics et rien n'est mis en oeuvre pour la filière bio, on peut s'interroger sur cet aspect et à titre d'exemple, les plans de soutien à la consommation pour la fouille de filière produits laitiers se chiffre à 20 millions d'euros et ce sont 175 millions d'euros qui ont été débloqués en 2022 pour se tenir la filière porcine. on peut se demander pourquoi ce différentiel de traitement. Le seul petit geste effectué par dans ce PDF a été le maintien du montant du fonds Avenir Bio. Le ministre de l'Agriculture a également annoncé hein. Il y a pas très longtemps en séance sur la mission Agriculture. D'accepter de financer un plan de communication donc on, on attend toujours cela mais sans moyens humains supplémentaires pour l'Agence Bio, chargée d'instruire les dossiers de fond d'Avenir Bio et de mener. Opération de communication, ces éléments qui reste insuffisant donc que peu de sens et ne seront pas véritablement opérants

Je ne sais pas si c'est un passage à vide mais enfin certaines difficultés les moyens sont maintenus sont même. Vous l'avez dit un peu augmenté par le Fonds bio, un certain nombre de productions. Aujourd'hui que soit fruits et légumes, beurre, farine, c'est entre moins 10 et moins 20% donc je pense que les. À ce stade les les moyens sont maintenus.--

après l'année 2023 en fonction de, de la manière dont ça va se passer pour éventuellement imaginer dans le prochain PLF venir en soutien, donc une demande de retrait pour ces amendements. Monsieur le Ministre même avis. Je mets aux voix ces amendements qui ont reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Ils ne sont pas adopté le 12 83. Monsieur le Ministre, c'est à vous.-- Oui, très rapidement, là aussi, il s'agit. D'une, de, d'ajustements qui sont fait cette fois-ci pour les plafonds d'emplois des opérateurs de l'État. Je vais rapidement nous augmentons de 4. ETP le plafond d'emplois de la mission cohésion des territoires au titre du transfert à l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, la une, c'était de la gestion du fonds pour une société numérique on avait ouvert les crédits en PLFR on a juste le plafond d'emplois en conséquence dans le PLF 23 il y a également une augmentation de 4 TP au ministère de la justice pour l'exécution du plan de charge de l'agence publique pour l'immobilier de la justice. J'ajoute également 3 ETP. Dans le cadre de la mission, contrôle de la circulation et du stationnement routiers à l'entaille. L'Agence nationale de traitement automatisé des infractions puisque il s'agit de mettre en gestion 5 nouvelles amendes forfaitaires délictuelles et le suivi de cette nouveau délit à la suite de leur forfaitisation et puis enfin le plafond d'emplois de l'office, l'Office français de l'immigration et l'intégration est augmenté de 20 ETP pour assurer le suivi et l'accompagnement des réfugiés ukrainiens.--

Qui est contre qui. S'abstient adopté 2 amendements identiques. Monsieur mais de vielles c'est vous qui défendez le 331 de la commission du développement durable. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre. Oui, cet amendement vise à augmenter les moyens humains du Conservatoire du littoral de 8 équivalents temps plein en 2023. Contre stagnation d'effectifs. Initialement prévu le Conservatoire du littoral est confronté depuis plusieurs années à une stagnation de son plafond d'emplois alors même que son domaine foncier. Ne cesse de croître au tire de sa mission, entre 2500 et 3500 hectares par an. Cet opérateur de l'État entretient dans tous les territoires littoraux des Liens très étroits avec les collectivités leurs élus qui gère une grande partie de son domaine. Il est un peu

Allez-y et vous reviendrez pour le suivant, monsieur Medvedev. Oui donc on, on l'a adopté à l'unanimité à la commission de l'aménagement du territoire et du moment durable. Il s'agit de résoudre le problème de VNF qui est victime de la contradiction entre deux trajectoires la trajectoire que lui fixe son contrat d'objectifs et de performance trajectoire de 3 milliards d'euros en faveur des infrastructures avec des objectifs ambitieux. Et par contre une trajectoire à la baisse de ses effectifs. Sur ces 3 dernières années. Une trajectoire à la baisse qui devrait se poursuivre en 2023 avec 40 TP en moins et donc cet amendement vise à en gros a assuré 40 TP ce qui garantit une stabilité entre 2023 et 2022. Six président requis les défendu merci qui est de l'avis de la commission. Une demande de retrait puisque. Le, l'amendement qui a été défendu dans la nuit de vendredi à samedi portait justement sur les amendes ma crédits les les 2 amendements qui ont été présentés ont été retirés, ce qui rendrait difficile en cas d'adoption, puisque si on adopté ces crédits, ça veut dire que ce serait prélevée sur le budget de VNF dont vous soulignez déjà qu'il est déficitaire. Je pense qu'il faut qu'on mette de la cohérence. Donc je, à un moment de retraite.-- Merci monsieur le ministre de ma vie je mets aux voix double avis défavorable qui est pour. Qui est contre

Non vous défendez votre amendement comme vous le son comme vous le souhaitez. Dans le renfort de 2023 des moyens du conservatoire permettra d'intervenir sur 3 champs prioritaires comme les rédactions des collectivités territoriales. De nouveaux projets de rester opérationnel d'écosystèmes terre-mer ou fragile ou fragilisées et donc sensibles aux changements climatiques renaturation de forêts incendiées résorption de charges littoral contribution à la recomposition spatiale. La flexibilité du trait de côte de nouveaux projets favorable la stratégie nationale des aires protégées pour reconquérir la biodiversité sur les futures zones de protection forte du Conservatoire Littoral. Et une action foncière efficiente pour contribuer à l'atteinte sous littoral de l'objectif ciblé du zéro artificialisation nette avec des chantiers de déconstruction permet réalisation et de renaturation. Aussi, afin de permettre aux conservateurs sur le littoral de poursuivre la tête du objectifs ambitieux fixés par l'État en matière de protection de sauvegarde de se passer du rôle. Il est proposé d'augmenter de 8 équivalents temps plein ses effectifs en 2023.

Ne cesse de croître. Cette augmentation du nombre d'emplois permettrait au conservatoire de de remplir au mieux ses missions en outre cet amendement permet de donner en partie les moyens à l'État et à ses structures de s'engager pleinement dans une transition écologique réussi et je crois que nous le souhaitons tous, donc j'espère que cet amendement. Aura un avis favorable. Merci nous prononcer. Six amendements identiques maintenant le 73 Madame Noël. Oui merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, il s'agit du même. Amendement qui les deux qui viennent d'être défendus précédemment, je demande de juste sept équivalents temps plein contre 8 précédemment. Merci.

d'augmenter de sept équivalents temps plein pour porter à 12 puisque il y a eu 5 TP qui ont été. Adoptées supplémentaire à l'Assemblée nationale, je voudrais dire que le conservatoire du littoral à des missions qui. Sont de plus en plus importante. Compte tenu de l'attention que nous portons à à à l'environnement mais aussi de la situation. Je vais citer quelques projets quand même la renaturation l'adaptation au changement climatique avec l'augmentation des niveaux de la mer la renaturation des forêts incendiées de résorption par exemple de décharge littoral ce sont tout un tas de missions supplémentaires qui prennent de plus en plus de temps donc. Le conservatoire du littoral a besoin de ses équivalents temps plein. On le voit dans beaucoup de services publics à partir du moment où on réduit

Hé bien, ça va être très simple effectivement le l'amendement de de repli si les sept n'était pas adopté, je vous propose au moins de d'accorder. Au Conservatoire du littoral 3 équivalents temps plein et donc, ce qui permettrait de d'amortir les difficultés qui sont considérables pour mener à bien l'émission de ce conservatoire. Je vous remercie madame la présidente. Vous avez. Par plusieurs fois appelé la tension sur les effectifs du Conservatoire du littoral. Ça a été dit par certains d'entre vous 5. Équivalents temps plein supplémentaires. Sont arrivés en création par le biais de l'article 49 3. Une des difficultés ou la principale difficulté. Que je vois à ces créations donc de 8 7 ou trois postes c'est qu'il n'y a pas de crédit pour accompagner ces créations de postes. comme tout à l'heure avec VNF. Ça veut dire que ça va être prélevé sur le budget du Conservatoire du littoral, dont vous dites qu'il est déjà. Un peu à flux tendu. Moi je propose 2 choses, la première c'est de regarder déjà ce que va donner. Le renfort des 5 équivalents temps plein supplémentaires. Il y aura toujours la possibilité après, en cours de gestion éventuellement d'imaginer un nouveau relèvement mais. au regard des prises de parole des uns des autres. Je je propose également que le ministre nous dise de quelle manière le gouvernement voit au regard de ses 5 postes créés. L'avenir sur l'année 2023. Pour ma part, ce sera une demande de retrait.-- Sur tous.-- D'accord. Monsieur le Ministre.-- Oui, évidemment on est très attaché à l'action du Conservatoire du. Littoral qui est au coeur de notre action pour la préservation du littoral. Français et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé dans le cadre du 49.3 sur le PLF. À l'Assemblée de relever déjà le plafond d'emplois. Je crois que c'était cinq c'est ça. ce qui témoigne encore une fois notre souhait de de le renforcer dans ses actions. Évidemment, on va continuer à le. Renforcer le fait d'avoir relevé de 5 ETP porte ainsi à 145 le nombre de TP du conservatoire autorisé en loi de finances, il pourra. S'appuyer également sur 20 ETP hors plafond qui sont prévues pour 2023. Donc pour ces raisons. Ça me semble satisfait et donc demande de retrait également. Oui merci madame la présidente. Donc moi je vais je vais maintenir les amendements parce que. Les 5 TP qui ont été adoptées à l'Assemblée nationale il on a bien trouvé les moyens de, de pour les pour pour les obtenir. Donc. Je garde les deux amendements les 7 ETP ou l'amendement de repli des 3 ETP. Je vous remercie. Merci. Monsieur Savoldelli.-- Oui madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues. Ben c'est le, c'est le point de départ de l'ouverture de nos travaux. Pour le rapporteur général demande de retrait pour le gouvernement satisfait.-- On parle de 5, nommé Les 120.000 ils sont là et 120.000 fonctionnaires vous avez-vous décidé de supprimer, ils sont là. Alors après il y a un jour à toi, à moi. Retrait lottini satisfaisant le ministre. Mais au final, moi je vais vous dire, je n'ai pas l'expertise nécessaire pour apprécier le nombre d'en d'emploi qu'il faut créer pour la la la surveillance du littoral mais moi j'ai confiance dans les collègues.-- Et là franchement c'est pas une demande pharaonique.

Bien je vais donc il n'y a pas d'autre explication de vote. Métro voit ces amendements, 224 et 11, 59 double avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Il est adopté. Ils sont adoptés et ils font donc tomber les amendements de repli. Bien entendu nous passons ensuite au 11 69. Monsieur Cosic. Merci madame la présidente. Donc c'est un amendement prison proposée par ma collègue Martine Filleul le respect du droit à l'information et la participation du public dans les débats relation des projets et des politiques ayant un impact sur l'environnement est fondamental.-- Nous sommes collectivement convaincus qu'associer les populations en amont, permet de bâtir des projets et des politiques publiques. Pertinentes qui s'insèrent dans le tissu social économique de nos territoires et in fine et de voir nos concitoyens s'approprier ce si. La concertation avec ces populations, on n'est pas accessoire, sortir de la logique de l'individu consommateur en privilégiant celle du citoyen acteur dans la vie de la cité est une nécessité aussi le le présent amendement propose de majorer le plafond d'emplois de 4 unités au sein de la commission nationale du débat public du débat public la CNDP afin d'augmenter ses moyens humains en vue, l'organisation des débats publics à venir liés aux énergies renouvelables et plus largement au choix démocratique liés à la plage des planification écologique. Quel est l'avis de la commission sur cet amendement. Une demande de de de retrait je moi je propose et j'en profite pour le dire au ministre, je propose qu'. Un état des lieux de des différentes. Instances qui sont en charge d'organiser le débat public de participer à la construction de, de l'opinion sur. Des sujets multiples et divers enfin tout ce qui est démarches participatives qu'on est un peu un état des lieux, parce que les organismes, les instances s'additionnent les unes aux autres, avec finalement une certaine difficulté à y voir vraiment clair. Une demande de retrait. Roche. La présidente, je je je voulais reprendre l'argument à la fois du rapporteur malgré qu'il ait pas donné d'avis favorable et celui qui a été présenté pour l'amendement de Madame de monsieur filleul de Madame Filleul en fait tout le mode met en place des politiques participatif partout parce que nous savons tous que c'est une nécessité absolue aujourd'hui de de de mettre en place ce type de politique et de trouver tous les moyens de faire participer les citoyens. Donc je pense qu'on ne peut pas ne pas avancer, faire un état des lieux. Certes je suis d'accord mais à un moment donné l'état des lieux lieux doit permettre aussi d'avancer en même temps donc je suis pour un état des lieux. Monsieur le rapporteur. Mais je suis aussi pour cet amendement parce qu'il faut commencer à avancer maintenant.-- Je vais donc mettre aux voix cet amendement qui a un double avis défavorable qui est pour.

Article 37. Ah le 11 68 2 amendements identiques Monsieur Féraud. Merci madame la présidente, je présente cet amendement du groupe socialiste, dont l'initiative revient à notre collègue Marie-Arlette Carlotti cet amendement concerne la métropole Aix- Marseille-Provence, et en particulier les relations financières entre la métropole et ses communes membres. Il fait suite à l'avis rendu par la chambre régionale des comptes, conformément à ce que prévoyait la loi 3DS de février dernier. Ah. Rapport sur. Le niveau des attributions de compensation, versée aux communes par la métropole et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans l'avis rendu cet été. La chambre régionale des comptes constate que la métropole à verser 631 millions d'euros d'attributions de compensation aux communes membres 2021 alors que la chambre évalue pour ce même exercice le montant de référence des attributions à 453 millions d'euros seulement. La chambre régionale des comptes souligne que cette. Surévaluation manifeste des attributions de de compensation nuit à l'équilibre budgétaire de la métropole réduit ses propres capacités d'investissement et se fait au détriment des communes pauvres et des territoires les plus fragiles socialement notre amendement prévoit donc une procédure pour encadrer un niveau des attributions de compensation de la métropole aux communes qui soit conforme aux charges transférées et qui permet d'instituer une dotation de solidarité communautaire pour réduire les disparités de ressources et de charges et les grandes inégalités de richesse entre les communes afin de les compenser il être accompagné de garanties qui vise. À respecter le principe de libre administration de chacune des communes dans le cadre de ses nouvelles, de nouvelles dispositions qu'il propose. Je vous remercie. Ou sur l'émission de de l'État dans le travail des collectivités et je les partage cependant surtout hélas je pense que cet amendement est nécessaire face à une situation de blocage dû à la fois à la situation locale et à l'écriture de la loi 3DS qui comme j'ai eu l'occasion de le dire s'est arrêté au milieu du gué. Certes, la question financière a en fait été posée avec la commode de de rapport auprès de la CRC sur les relations financières entre la métropole et les communes le 1er rapport a été remis en octobre, il a mis en évidence. Près de 180 millions d'euros de versements appelé du et versement qui aurait été fait aux dépens in fine et de la métropole. Voilà où nous en sommes constat sans appel d'une métropole n'ayant pas les moyens d'agir et de communes dans les flux financiers perçus ne relève pas de la stricte neutralité des transferts de compétences, il faut que tout le monde le sache. Et nous voilà dans une situation très très fragile. Le rapport existe. Il a été demandé par le Sénat et la loi 3DS. Il se pourrait que rien ne change. La métropole doit retrouver des moyens de ses compétences, celle de porter de nombreux projets à une échelle pertinente. Les communes doivent retrouver les moyens d'agir dans leurs compétences. Cet amendement va dans ce sens, le sens d'une répartition juste équilibrée progressive les crêtes sans prise en compte et et l'amendement ne prévoit pas la remise en cause de l'ensemble de ses 178 millions a dû, il prévoit seulement qu'au moins 50% soit redirigé vers les besoins réels à la fois des communes et de la métropole, il limite les impacts sur les communes en limitant la variation pour les Budgets des communes jusqu'ici bénéficiaire et le tout est lissé sur 4 ans. J'entends les réflexions sur laisser le temps à la concertation des acteurs locaux. Mais jusqu'à quand.-- Depuis plus d'un an, j'en ai alerté préfet Premier ministre-président de la République et président de la métropole cette métropole mal n'est fait l'objet de réflexions quasi annuelle et les changements acté ne sont que les prémices d'amélioration durable de son action au moment où l'État met en oeuvre un projet Marseille en grand la métropole et la commune de Marseille doivent retrouver des rapports financiers apaisée, le temps est à l'action et si j'avais à temps espéré que les communes et la métropole devant l'évidence parviennent à une sortie de satisfaits

profite pas à nos territoires et ne profite pas à nos communes.--

à côté et en plus de ce que vous avez évoqué sur le rapport de la chambre régionale des comptes, moi je veux. Peut être abordé plusieurs points qui m'amène. D'ores et déjà à rendre un avis défavorable. Tout d'abord en en remettant en cause. Le le le le. Fonctionnement actuel qui d'ailleurs. Est intégré dans les Budgets par les communes, on risque de fragiliser en tous les cas, les choix à venir et notamment d'investissements de certaines communes. Deuxièmement, je rappelle qu'un article du code général. Prévoit 4 types de procédures de révision de l'attribution de compensation. C'est soit la révision libre avec accord entre le PC et ses communes membres soit une révision lié à de nouveaux transferts de charges soit une révision unilatérale, sans accord entre le PC et les communes membres soit enfin une révision individualisé avec un accord entre le PCI et une majorité et une majorité qualifiée des communes membres. Je crois que c'est très important de se tenir à un de ces quatre cas troisièmement concernant la DC la dotation de solidarité communautaire. Elle était effectivement obligatoire pour les métropoles, même s'il est vrai qu'elle n'est que. Peut être symbolique relativement au sein de la métropole Aix-Marseille. Mais j'ajouterai enfin que, une fois ces constats faits. Il n'appartient pas, en tous les cas. Dans la libre administration des collectivités locales à une assemblée parlementaire de décider pour le compte d'assemblées locales qui ont leurs propres modalités de fonctionnement. Je crois que nous devons faire attention, et de ce que je crois comprendre sur les différentes sensibilités de l'échiquier politique. Il y a loin d'avoir une unanimité, raison de plus pour que dans notre assemblée. Nous restions prudents.-- d'une part de mettre en place une révision des attributions de compensation permettant, sur la base du rapport de la chambre régionale des comptes de PACA de revoir les montants versés aux communes, et d'autre part hein prévoit que par délibération une dotation de solidarité communautaire est institué égal aux 2 tiers du montant de la baisse des attributions de compensation. En cas d'absence de délibération. L'amendement prévoit également que le préfet saisit la chambre régionale des comptes pour fixer le montant des attributions de compensation et arrête la dotation de solidarité communautaire. Moi je veux rappeler 2 choses, d'abord la loi relative à la différenciation la loi 3DS disposer avec les élus locaux devaient tirer les conséquences de la vie de la chambre régionale des comptes sur les flux financiers entre la métropole et ses communes dans un délai. De deux mois après la communication de la vie. vie. 2ème, chose que je veux souligner c'est que 3 mois plus de 3 mois après la communication de la vie et alors que celui-ci a été rendu publique aucune initiative forte n'a été prise par les élus du territoire pour. Réviser les. Attributions de compensation. Instituer une dotation de solidarité communautaire et que donc la mesure qui est proposée par ces amendements, elle permet à une chose, c'est d'avancer et qu'on a besoin d'avancer pour Marseille, pour la métropole pour les Marseillais et dans le cadre du plan Marseille en grand, qui a été porté par le président de la République au bénéfice des Marseillais et donc pour ces raisons je donne un avis favorable à ces amendements.--

Il est frappé d'inconstitutionnalité puisque le rapporteur là l'a très bien dit, c'est la libre administration des collectivités territoriales et la que fait le législateur,

J'aurais voulu ne pas, ne jamais prendre la parole sur cet amendement, le 2ème aspect. Relisez bien l'amendement c'est technique du rabot. C'est-à-dire une ville comme Salon-de-Provence je prends juste cette ville dans le rapport de la chambre régionale des comptes. Ces 6 millions d'euros en 4 ans d'efforts sur son budget de fonctionnement. Juste 6 millions d'euros. Ça veut dire clairement un déséquilibre financier criant dans 4 années en fait on va appauvrir l'ensemble des communes au bénéfice de la ville centre. On parle de péréquation. Mais mes chers amis, la péréquation. Ce n'est pas la technique du rabot, c'est de prendre aux plus riches pour. Déverser aux plus pauvres. C'est ça la péréquation à travers la dotation de solidarité communautaire. C'est la véritable. Péréquation. Là aujourd'hui votre amendement ne propose pas ça. Il propose d'appauvrir tout le monde au profit de la commune sans, encore une fois il y a des charges de centralité, il y a des ressources qu'on pouvait aller chercher on avait présenté avec le sénateur Ben Haroche. La solution du versement mobilité est le déplafonnement ça nous a été balayé d'un revers de main par le gouvernement et maintenant le gouvernement ce même gouvernement vient nous dire attention il y a le plan Marseille, Marseille en grand à mettre en oeuvre, c'est pour ça que je, j'émets un avis défavorable.-- Il n'y a pas d'autres explications de vote, Monsieur Bénard Roche. bien sûr Stéphane Le Rudulier a défendu avec brillamment sa position. Cela étant dit, la partage pas, ne serait-ce pas vraiment une politique du rabot parce que il y a quand même des normes fixées avec des maximums autorisés enfin l'amendement effectivement faut bien lire et donc il faut lire tous ces articles dans l'amendement. En fait pourquoi cet amendement. C'est vraiment le reflet d'un espoir et d'un échec. Les chèques c'est de n'avoir pas dès la loi 3DS organiser les conséquences du rapport que remettrait la CRC dans chacun d'entre nous, y compris dans les Bouches-du-Rhône et surtout dans les Bouches-du-Rhône savait qu'elle allait être la teneur parce que personne ne se fait d'illusions. Soyons clairs, l'échec de la prise en compte en même temps, des besoins financiers conséquents de la métropole pour être à la hauteur de l'échelle de ces projets et la réalité du besoin de solidarité entre communes au sein de la métropole pour donner tout sans sauce. Ah au au sens au destin commun métropolitain. Ce qui est quand même important alors qu'on va définir l'intérêt métropolitain. Mais cet espoir qui a été co-construit avec des élus locaux, des parlementaires et le gouvernement depuis longue date peut voir enfin un équilibre plus juste des relations financières l'espoir avec la mobilisation d'ailleurs sur la même position non seulement de nos collègues socialistes dans la sénatrice des Bouches-du-Rhône Marie-Arlette Carlotti mais aussi du du sénateur des Bouches-du-Rhône Jérémy Bacchi. L'amendement a eu l'effet escompté. D'ailleurs, jeudi, réunion du conseil métropolitain des mères et comme par hasard sur la table une proposition est faite jeudi soir après le dépôt de l'abonnement et la position du maire de Marseille Benoît Payan, qui le défend. Prévu initialement comme repli en cas de non-accord local. D'accord. Trop tardive, voire de statu quo indécent après la parution du rapport de la CRC, les acteurs locaux à jouer le jeu, ils ont pris leurs responsabilités et les baronnies d'hier ont laissé place à des discussions sérieuses, je l'avoue. Des avancées réelles, sur des je suis d'accord avec vous et un engagement de répartition des moyens entre une métropole qui a besoin de ressources pour financer ses projets et des communes qui sent la solidarité ne peuvent appartenir au destin commun du territoire ni porter leurs compétences propres que la loi 3DS Laurent ce n'est qu'un début mai à cette heure je ne sais pas quelle heure il est, aujourd'hui, rien n'a été acté, rien n'a été écrit, rien n'a été signé jeudi encore confirmation, vous savez qu'Emmanuel Macron était à ma à Aix aujourd'hui et les discussions ont eu beau très autre Emmanuel Macron Martine Vassal Benoît Paillaugue, vous le savez tous, aussi bien que moi, surtout ceux qui sort des Bouches-du-Rhône.

Assez bien coordonnées. Si j'ai tout compris, un peu du gouvernement et puis on essaie de trouver. Des accords locaux. Ce que je comprends quand même c'est qu'il semblerait que les choses bougent. Et je vais vous dire, je crois qu'ici. Si ça doit bouger c'est localement que ça allait bouger.-- Puisque. Je me suis même laissé dire que. Ça aurait l'Avantage de contraindre un peu plus vite, les acteurs locaux à trouver une solution. Et à se réunir, mais je pense qu'ils n'ont pas besoin enfin je, je le redis libre libre administration des collectivités locales. On le dit. Non mais moi je suis pas là depuis 10 ans. Je dis simplement, quelle est la situation aujourd'hui. Donc qu'on laisse la libre administration des collectivités locales. En plus on va se le dire les majorités ont changé. Les équipes également. C'est en train de bouger, ben faisons confiance et je crois comprendre que vous faites partie de ces acteurs locaux. Ben c'est le moment de faire avancer le dispositif mais je ne crois pas qu'il faille effectivement mettre trop de verticalité ou de décisions parisiennes pour imposer à la métropole Aix-Marseille qui mérite quand même de pouvoir choisir souverainement par elles-mêmes.-- Merci. Alors avant de procéder au vote. Je répondais à une presque question posée même collègue ben arrange, ce qui était je ne sais pas quelle heure il est. Alors il est 22h 16 et il reste sans ces amendements examinés. amendement qui a reçu ces deux amendements identiques, qui ont reçu un avis défavorable de la commission est favorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre Ils ne sont pas adopté. 3 amendements identiques de suppression madame Vermeillet.-- Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, l'article 109 de la loi de finances pour 2022, rendait obligatoire le reversement de tout ou partie de la taxe d'aménagement entre entre communes et EPCI en fonction des charges d'équipements publics assumées par chacune des collectivités. Lors de l'examen du second projet de loi de finances rectificative pour 2022, le groupe Union centriste a fait adopter un amendement visant à revenir à la situation antérieure à celle créée par cet article 109 de la loi de finances 2022 et par conséquent sur l'obligation pour les communes de délibérer sur l'affectation d'une fraction du produit de la taxe d'aménagement à leur EPCI. Cette mesure a été conservé dans le texte final de la CMP qui est parvenu à un accord par coordination et afin de garantir le retour pérenne à la situation antérieure. Cet amendement propose de supprimer l'article 37 du PLF 2023 devenue sans objet, merci.-- merci.-- Rapporteur général défendu. Monsieur ça vole. Oui merci madame la présidente ce le Ministre, mes chers collègues. Ça a été bien expliqué mais la réforme de la répartition de la taxe d'aménagement. L à chambouler un équilibre. Et l'équilibre qui a été trouvé entre les communes et les EPCI.-- La date butoir du premier octobre 2022 pour délibérer de la répartition a remis le sujet sur la table ah permettant à tous les élus locaux de constate à niveau, à quel point cette réforme constituait un contresens.-- Et là j'ai je prendrai appui pour mon groupe à ce qui a été dit par l'Association des maires ruraux de France. Les mots sont justes.-- Je cite, ni le fondement même de la Namik de coopération intercommunale.-- Cette réforme elle ni le fondement même de la dynamique de coopération. Selon les équipements intercommunaux que la commune accueille alors elle pourra déterminer si elle entend renverser ou tout ou partie du produit de sa taxe d'aménagement. Et donc l'aspect injuste de cette réforme menée d'ailleurs sans concertation se concrétise lorsque au simple constat que toutes les communes doivent reverser un taux identique alors que les équipements intercommunaux sont de très peu, voire très voire très peu ou voire même très très peu sur leur commune. Donc les modalités de reversements sont d'autant plus laborieuse que les modalités de calcul sont floues et cette obligation délibéré ressemblaient fâcheusement à une nouvelle injonction gouvernementale s'inscrivant dans un lent mais pas moins violent mouvement de tutelle nisation des collectivités locales. J'ai pu lire même des élus, des maires. Dans ça. Notamment les maires de petites villes.-- Parler d'une forme d'infantilisation des mères donc pourquoi décider au détour d'une loi de finances que les communes qui subissent d'ailleurs l'envolée des prix de l'énergie. L'envolée des denrées minime enterre ont perdu la taxe d'habitation devraient reverser plus 10% du produit de leur taxe d'aménagement.-- Je pense qu'il faut donc aller à la suppression, merci.-- Je mets donc aux voix ces amendements qui ont reçu un avis favorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Ils sont adoptés et font donc tomber. Tout jusqu'à l'article et nous passons aux 37. pardon monsieur rapport général de la parole.-- Je vous donne la parole, avant les amendements. Si madame la présidente, je veux dire quelques mots. Ce qu'il y a beaucoup d'amendements relatifs à la répartition du produit diffère faire donc on va aborder ces amendements. Qui finalement pose la question de la répartition du produit diffère entre les collectivités. Je rappelle que l'IFER est une taxe qui vise à intéresser fiscalement les collectivités à l'implantation de certaines installations sur leur territoire. À l'exemple par exemple pour ce qui nous concerne aujourd'hui des éoliennes ou des centrales photovoltaïque ou hydraulique. Ces règles. Les modalités de répartition de son produit entre communes, EPCI et départements peuvent varier à ce actuellement selon la nature des installations tous ces amendements pour cibles même objectif renforcer la part perçue par les communes afin de les inciter à s'engager davantage dans les projets. La loi de finances initiale pour 2019 a fait d'ailleurs à premier pas en la matière en transférant 20% du produit diffère sur les éoliennes nouvellement installés afin de parvenir à la répartition suivante, à la répartition suivante, 20% pour la commune, 50% pour le PCI, 30% pour le département. Je rappelle que la commission des finances, il était défavorable car la répartition éolien lui paraissait conforme à la répartition des compétences entre chaque échelon. La seconde loi de finances rectificative pour 2022 adopté la semaine dernière, suite à un accord en CMP prévoit un alignement de l'IFER photovoltaïque en transférant de nouveau 20% du produit du département vers les communes au titre des centrales installées à compter de 2023 on arrive donc à une même répartition 20 50, 30 qui satisfait d'ores et déjà plusieurs des amendements déposés. Dès lors, il ne semble pas opportun de bouleverser à nouveau c'est tout récent équilibre que nous avons posée, d'autant plus que nous travaillons et je veux le dire tout de suite ici à enveloppe constante et donc tout renforcement de la part communale se fait ou se ferait au détriment des autres échelons pour cette raison je demanderai donc le retrait de tous les amendements à part de. Un premier qui. Compte tenu du nombre d'amendements sur le sujet, je proposerai de m'en remettre à la sagesse de notre assemblée sur l'amendement 136 du sénateur Rapin, qui vise à ce que les communes perçoivent 20% de l'IFER éolien y compris au des installations datant d'avant 2019. Je me permets néanmoins d'attirer notre attention sur le fait qu'une telle mesure entraînerait ou entraînera une perte sèche d'assiette fiscale pour les intercommunalités. Sans avoir d'effet incitatif puisque les éoliennes sont déjà installés ensuite et enfin je solliciterai l'avis du Gouvernement sur l'amendement du sénateur Maurey le 171 relatif cette fois au partage du produit diffère entre communes limitrophes lorsqu'une éolienne est situé à proximité immédiate pour ne pas dire à la frontière entre des périmètres territoriaux en m'interrogeant notamment sur la faisabilité technique du dispositif et les risques éventuels qu'un tel amendement pourrait provoquer en terme si j'ose dire de saupoudrage. Merci. Nous allons donc maintenant examiner les amendements auxquels le rapporteur a donné déjà son avis. Très bien. Et le 12 04. Monsieur le Président requis. Merci madame la présidente, monsieur le 1000 chers collègues le présent amendement vise à permettre aux territoires accueillant parc solaire de pouvoir bénéficier des retombées positives liées au dynamisme économique induit par le débordement des énergies renouvelables afin de renforcer la la l'acceptabilité locale des installations. Pour ce faire, il est proposé de prévoir une part de 50%, de lui faire relatives aux hein sergent photovoltaïque soit attribués à la commune 32%. Ah le PC. Et 20% départements y compris en cas de renouvellement du installations existantes par délibération la commune ne peut également permettre au bloc communal se substituer pour une facture de l'hiver qu'elle perçoit cessent de justifiant la décision se justifie par ailleurs par le besoin pour l'ensemble des communes portant des projets solaires sur leur territoire de justifier d'une recette directe et pérenne.-- Madame Noël pour le 96. dans l'acceptation des projets des populations locales ou encore dans la garantie des conditions permettant à ses installations de fonctionner correctement. En effet, un lecteur actuel. La loi prévoit que l'IFER à laquelle sont assujettis ces installations est en très grande majorité reversée aux départements et aux intercommunalités qui ne jouent pourtant aucun rôle dans la concrétisation de ces projets et sans garantie de retour sur le territoire communal en terme de service. Le présent amendement instaure donc un partage plus juste du produit de l'IFER relatives aux éoliennes et aux centrales photovoltaïque photovoltaïque pardon en réduisant à 35% la part reversée aux intercommunalités au profit des communes.

Alors la présidente. C'était un alignement de l'IFER. Photovoltaïques sur les faire éolien, c'est ce que vient de dire le rapporteur général. Il est donc satisfait. Je vous remercie. Merci madame Vermeillet pour le 54. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, monsieur le rapporteur général. J'ai écouté les explications du rapporteur général donc mon amendement propose que. Les communes qui accueillent des installations photovoltaïques perçoit 20% de l'IFER. Simplement, le rapporteur général explique que il y a un avis favorable pour les installations à compter de 2023 et notre amendement prévoit que ce soit pour l'ensemble. C'est-à-dire que ça concerne les installations existantes et je trouve ça très juste, je l'ai déjà défendu. Lors du du PLFR de tout simplement parce que les communes qui ont déjà des installations, photos. Photovoltaïque, elles ont été pionnière et je trouverais ça très injuste qu'on leur dise ben vous avez fait ça trop tôt. Donc vous n'aurez aucun bénéfice du partage de lui faire et si je suis d'accord avec l'amendement du sénateur Rapin, sur le fait que on revienne sur l'éolien sur des installations antérieurs à 2019, il s'exile. Il s'agit exactement de la même chose je trouve que le photovoltaïque. Il doit aussi bénéficier aux installations antérieurs. Donc pour moi c'est une mesure de justice et j'espère que. On accordera à l'ensemble de ceux des communes qui ont. Été pionnière et qui ont osé se lancer dans, dans des investissements de cette nature, de pouvoir bénéficier elle aussi de l'IFER. Photovoltaïque merci. Oui, donc on a bien compris que sur le principe. Les choses avaient avancé sur le 20 50 30 20 % pour les communes, 50% pour les EPCI et 30% pour les départements. Nous notre amendement propose de ne pas revenir avant 2019 mais quand même de partir du 1er janvier 2019, ce qui correspond aussi à des installations assez mature dans dans le développement du photovoltaïque. Donc j'ai l'impression que le débat c'est 2023, 2019 ou avant 2019. Donc là il y a quand même encore un peu de débat.-- merci madame la présidente. Donc c'est un amendement proposé par mon collègue Losec. Qui propose d'instaurer un partage plus juste de l'IFER relatives aux centrales photovoltaïques au niveau du bloc communal en réduisant de 50 à 30% tout au plus la part reversée aux intercommunalités ont AFP U et permet ainsi d'établir à 20% au minimum la part reversée aux communes.-- Oui madame la présidente, monsieur j'ai plus grand chose à dire puisqu'il a été des plus ou moins défendu par le rapporteur et puis je remercie Sylvie Vermeillet. D'avoir défendu mon amendement mais le principe, c'est effectivement de ne pas l'analyser les communes. Qui ont qui ont implanté des des éoliennes sur leur territoire avant le 1er janvier 2019 et de leur permettre de participer aussi à ce à cette réversion de la partie. d'un. Il s'agit de faire évoluer la répartition, de les faire pour intéresser les communes au. Voltaïque photovoltaïque prenant en considération que beaucoup sont des communes rurales et qu'il faut bien et c'est évidemment les encourager dans cette voie là en ayant des projets qui soient attractifs incitatifs au même titre que l'éolien.-- Cet amendement d'Hervé Maurey propose de réserver son le produit. De l'hiver, à part égale entre la commune 50% et le PCI 50% auquel elle appartient. Le 94, madame Noël défendu. Le. 171 madame Vermeillet. Défendu. Président OK 12 07 défendu. Quel est l'avis du gouvernement sur ces amendements.-- Merci madame la présidente. Je donne un avis défavorable sur l'ensemble des amendements et je vais me concentrer pour. Les motivations sur les deux amendements pour lesquels le rapporteur général a donner soit un avis de sagesse le 136 soit demander l'avis du gouvernement pour le 171. Moi je veux d'abord rappeler à titre liminaire que il y a eu une réforme sur l'IFER éolien en 2019. Et que notre souhait, ça n'est pas dans bousculer les équilibres, nous avons repris la philosophie et vous avez repris d'une certaine manière la philosophie de cette réforme pour l'IFER photovoltaïque dans le cadre du PLFR puisqu'à la suite de la CMP, une mesure a été adoptée dans le PLFR, qui s'inscrit finalement dans la même philosophie que la réforme de 2019 sur l'IFER faire Sur l'amendement de Monsieur. Raffarin moi je je. Je veux rappeler que quand on a modifié la répartition. Ça a toujours été fait pour l'avenir. Là en l'occurrence ça reviendrait à à changer pour le passé et pour ce qu'il a déjà été. Installé. Or nous ce qu'on souhaite c'est éviter de faire perdre des ressources au département je je l'assume. Et la 2ème chose c'est que ces ces demandes. Enfin les demandes de, de revoir la répartition qui avait été fait elles étaient motivées avant tout dans une logique incitative pour inciter à l'installation d'équipements. Or si on change les règles a posteriori pour le passer, il y a plus cet enjeu incitatif puisque par définition les installations ont déjà été ont déjà pour ces raisons-là défavorable sur le 160 et 11. Je comprends la philosophie de l'amendement de monsieur Moret qui consiste à dire il y a des communes qui n'accueille pas sur leur territoire. Un équipement. C'est sur la commune d'à côté. La commune. Qui ne l'a pas sur son territoire à elle peut se prendre entre guillemets une partie de la nuisance visuelle ou autre, sans pour autant bénéficier de la ressource qui va avec l'installation de l'équipement. J'entends parfaitement ce qui enfin la philosophie. Moi je veux rappeler hein que quand vous avez un équipement qui est à cheval sur 2 communes, c'est évidemment à la ressource évidemment reversé au prorata pour les différentes communes et de surtout que la part qui aujourd'hui versée aux communes par rapport à l'Interco est quand même assez faible. Et que donc ma crainte, c'est que si on la réduit encore à la fin ça laisse assez peu de caractère incitatif pour une commune pour installer des équipements et que par ailleurs il y a une part importante qui va à l'Interco. C'est aussi dans une logique que l'intercommunalité puisse en reverser une partie, ou en tout cas compenser pour des communes qui seraient affectés par l'équipement sans bénéficie directement de la ressource. Donc pour cet avis également défavorable, 160 et 11.-- Merci je vais donc. Madame Vermeillet.

même avant 2019 ça vous êtes en train de me dire par rapport à l'amendement de Monsieur Rapin que toutes celles qui ont eu des installations avant 2019 pour de l'éolien et moi je parle aussi pour le photovoltaïque. Bah du coup elles elles peuvent avoir les nuisances et aucun bénéfice. Donc je comprends pas et pour moi c'est celles qui ont des nuisances et ben elles ont un peu de bénéfice et si on on n'accepte pas cette idée là hé ben on ne développera plus rien.-- Oui merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, moi je. L'tout d'abord me me ranger à l'avis du rapporteur général qui a rappelé effectivement l'harmonisation sur laquelle nous avons déjà avancé sur les les on peut aller faire entre le photovoltaïque et et et l'éolien qui me semble être effectivement un, un bon équilibre et sur lequel il faut sans doute s'arrêter. Ce qui me semble être la proposition retenue par ailleurs moi j'entends les les remarque temporelle hein c'est-à-dire que par rapport à ses et ces ces équipements qui sont aujourd'hui taxable je ne vois pas pourquoi ne seraient taxés que ceux qui seraient mises en place à partir de 2023 et donc je rejoins plutôt la vie que c'est c'est l'équipement qui mérite d'être taxés et non pas la date à partir de, du, duquel celui-ci est implanté et puis je voulais juste profiter une seconde De la parole sur cet amendement pour faire une observation sur un autre sujet qui aujourd'hui ne fait pas l'objet d'une répartition équitable dans le bloc communal sont les postes de transformation électrique qui sont intégralement à 100% diffère pour l'intercommunalité alors que souvent pour les communes, c'est un poste de charges, notamment pour la desserte en terme de voirie communale. Donc c'est une sorte d'appel pour examiner aussi une harmonisation à ce à ce niveau-là, je vous remercie. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Vous avez vu nos, notre groupe n'a pas déposé d'amendement et va participer au vote. Évidemment, la fiscalité des des éoliennes et l'implantation d'énergies renouvelables, en général c'est un enjeu de développement de l'éolien.-- Mais je vous avoue que.-- Quand on regarde ce qui vient de se dérouler là. La baisse des impôts de production.-- Qui va quand même beaucoup impacté les 3 niveaux de collectivités. Le retour de l'inflation.-- Qui pèse sur les achats et la hausse et on y on ni maire ni ajoute pour l'année là qui va être Yoanna, les plaines avec la hausse du point d'indice des des fonctionnaires, ça crée quand même une tension terrible pour toutes les collectivités à tous les niveaux.-- Je vous avoue que on on aura des votes différents suivant les amendements.-- Mais voilà, on n'en a pas déposé parce que nous on pensait que là c'était vraiment pas le moment de de mètres sans le vouloir forcément en cherchant des ajustements. Mais de, de Maistre les échelons territoriaux en opposition. Voilà, je vous le dis c'est c'est une position, ce qui va nous amener à voter pour s'abstenir ou contre. Mais voilà, on pense que c'est des amendements qui sont à la marge et qui ont quand même le problème de mettre en opposition les 3 niveaux de collectivités dans la clé de répartition de Bien s'il n'y a plus de d'explication de vote je vais mettre aux voix ces amendements. D'abord je vais mettent successivement neuf amendements qui ont tous reçu un double avis défavorable jusqu'au 136 de notre collègue Rapin. Le 12 04 qui est pour.

Qui est contre. Qui savent, ce n'est pas adopté le 725 et pour. Qui compte qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Je mets aux voix le 136 qui a reçu un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du gouvernement qui est pour.

Qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Le ce 94. Qui est pour.-- Qui contrôle qui s'abstient pas adopté acheter. Le 171. Monsieur le rapporteur. Vous demandez l'avis du gouvernement. Vous vous ranger à l'avis du gouvernement, donc double avis défavorable. Qui est pour.

Oui madame la présidente, monsieur le ministre, il s'agit d'un amendement déposé par mon collègue Cédric Vial qui concerne les EPCI à fiscalité additionnelle. La dotation de solidarité communautaire qui permettait de répartir en fonction de critères librement déterminés dans les statuts de l'intercommunalité a été remise en cause par le vote du PLF 2021 et depuis il n'est plus possible de le faire. De la même manière ces EPCI à fiscalité. Additionnelle dont donc plus aucun nous outil souple afin de procéder à des reversements de fiscalité à leur communes membres. Ce qui pourrait parfois permettent de débloquer un certain nombre de situations sur des sujets de fiscalité ou de rétrocession de compétences. C'est pourquoi cet amendement propose de mettre de à fiscalité additionnelle d'instituer des reversements de fiscalité aux communes facultative dans le cadre d'accord local entre EPCI et commune. Je précise que cet amendement a été travailler en lien avec l'AMF merci. Le 628 il est défendu monsieur Féraud. Et défendu merci quel l'avis de la commission.-- Alors sur ce dispositif donc de la dotation de solidarité communautaire. Effectivement c'est un dispositif qui a été modifié par la loi de finances de 2020. Ça a été également rappeler les règles applicables aux EPCI. Ciel unique ou à fiscalité additionnelle sont désormais unifiés. 7 décès et donc facultative pour les communautés d'agglomération et pour les communautés de communes. Elle est obligatoire pour les communautés urbaines. Cela signifie donc que les EPCI à fiscalité additionnelle peuvent mettre en place une décès et surtout si la plupart des communautés de communes applique en principe la fiscalité additionnelle. Elles peuvent tout tout à fait opter pour la fiscalité professionnelle unique un avis défavorable.-- Ils seront même avis. Je vais donc mettre aux voix c'est. 2 amendements identiques qui ont reçu un double avis défavorable qui est pour.

Ces syndicats mettent en 2 des actions et des projets en matière de transition énergétique de rénovation thermique des bâtiments publics communaux de développement des énergies renouvelables pour le compte des communes en toute logique ces syndicats devraient être éligible à la déciles dont le but est d'aider les collectivités territoriales à financer les projets favoriser en favorisant la transition énergétique. Ces syndicats peuvent intervenir que maître d'ouvrage de. De projets d'énergies renouvelables d'éclairage public en lieu et place des communes pour le compte de ces dernières. Or, ils ne peuvent percevoir d'aide au titre de la décile et les communes non plus puisqu'elles ont transféré leurs compétences. Pour toutes ces raisons, les auteurs de l'amendement estime que Cédric des syndicats devraient être éligible à la déciles pour mener à bien les projets de modernisation du parc d'éclairage public des collectivités.-- Merci, qui est de l'avis de la commission.-- C'est un avis défavorable. J'ai compris que c'était un amendement d'appel je veux rappeler d'abord que ces syndicats ou un mode de financement propre qu'ils perçoivent des recettes, notamment de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, la contribution des communes et également les redevances de concessions en fonctionnement et je rappelle enfin ce qui n'est pas rien, qu'ils disent que c'est même. Comment dirais-je, structure dispose en investissements des subventions du face et ce qui ne laisse pas ses structures sans moyens donc je leur ai dit un avis défavorable.-- Monsieur le Ministre, ma, ma vie. Je mais on voit qu'il est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il n'est pas adopté le 11 44, monsieur Cozic. Merci madame la présidente. Donc c'est un amendement que propose ma collègue sénatrice de la Charente Nicole Bonnefoy le présent amendement a pour objet de sécuriser les conventions de subventions conclu en matière d'aménagement. Numérique du territoire des projets de réseaux d'initiative publique. En effet, cet amendement est essentielle pour permettre de financer le déploiement du très haut débit. Dans les territoires concernés par une défaillance de montage institutionnel que la DGCL a identifié dans un certain nombre de départements ainsi pour le département de la Charente, la problématique rencontrée vient de l'illégalité dénoncée par la chambre régionale des comptes de la convention tripartite entre les et PCI le Syndicat départemental d'électricité et de gaz et le syndicat numérique qui pose un problème de financement en cascade.-- Si cette situation restait inchangé. Il y a un risque de bloquer des investissements pourtant budgétés par les collectivités. Rien que pour la Charente. Ils sont estimés à près de 30 millions d'euros et d'arrêter du même coup l'ensemble des travaux de raccordement. L'aménagement numérique du territoire est une priorité pour les départements à forte dominante rurale encore marqué par des zones blanches à l'heure où la numérisation des services publics se généralise tout ralentissement du très haut débit sera facteur de renforcement des inégalités territoriales.-- Pour résoudre ce blocage de nature purement administratif. Cet amendement permet de mettre en conformité le montage juridique et comptable du très haut débit. Cette solution repose sur une simplification du montage en donnant la possibilité aux EPCI de verser une subvention directement aux syndicats numérique en qualité de porteurs du projet de rip FTP FTTH départemental.-- Preuve de la pertinence de ce dispositif la Vicat soutient cet, cet amendement qui répond à des problématiques locales urgente et sécurise le financement du réseau fibré. Indispensable à nos concitoyens pour garantir l'égalité des territoires. ce sera une une demande de retrait. Quelques éléments d'explication, d'abord il peut être fait usage de fonds de concours dans quelques cas dérogatoires qui sont d'ailleurs précisément défini par la loi dont l'un d'ailleurs concerne l'établissement des réseaux publics de communication électronique par un syndicat mixte. Cet amendement. Risque de poser des difficultés juridiques liées notamment à la mise en place d'un fonds de concours. Nécessaires à la perception de cette subvention, la mise en place de fonds de concours est en effet strictement encadré par le droit et la jurisprudence, c'est notamment la cour administrative de Lyon. Qui a rendu un arrêt il y a quelques années et il n'est pas certain que cet amendement serait conforme à cette jurisprudence. J'ai bien entendu néanmoins. Le cas spécifique du département de la Charente. Donc j'imagine que Monsieur le Ministre, vous avez précisément sur sur ce cas si les unique des éléments de réponse, mais une demande de retrait.-- Oui. Même avis pour les mêmes raisons exprimé par le rapporteur. Le rapporteur général parce que l'amendement ouvre une dérogation au principe de spécialité qui régit l'exercice de leurs compétences par les EPCI et que cette dérogation ne nous sommes pas utile dans la mesure où le cadre relatif au financement de la compétence réseau numérique dont on parle ici apparaît comme susceptible d'offrir une solution ou. Acteur. Moi je suis prêt à ce qu'on regarde, je ne sais pas s'il y avait eu des rencontre peut être au niveau du cabinet de mon collègue Christophe Béchu. Ou de madame Cayeux sur le sujet pour regarder s'il y a des situations spécifiques. Ou. S'il y a des suites judiciaires. S'il y a un sujet spécifique, on peut regarder pour la Charente. Moi je n'en ai pas connaissance personnellement mais je pense qu'on peut regarder s'il y a un sujet spécifique sur le territoire de la Charente, mais en tout cas, il nous semble pas nécessaire de revenir et d'ouvrir une forme de de dérogations sur ce principe, comme l'a dit le rapporteur général. Si c'est pour un cas particulier qu'on doit pouvoir régler d'autres façons j'espère mais je vois que Monsieur chaise à l'air aussi motivés pour s'exprimer sur le sujet.-- je voudrais intervenir tout d'abord parce que j'ai été interpellé en tant que président d'AVIC, mais aussi pour dire que moi je vais soutenir cet amendement pourquoi parce que ça fait plus d'un an qu'on essaye de trouver des solutions et que aujourd'hui on se trouve. Dans dans une impasse qui fait que la. Le département de la Charente, risque de perdre plusieurs années dans le déploiement de son réseau fibre optique. Je crois qu'on a tous une volonté commune et le gouvernement dans lequel vous êtes en, en particulier pour faire en sorte que le déploiement de la fibre optique sur le territoire national se fasse dans les meilleures conditions. Eh bien en Charente si on ne trouve pas une solution, on va bloquer tous les investissements. Ça fait encore une fois. Plus d'un an, vraiment qu'on ait recherché auprès de la DGCL auprès de tous les acteurs pour trouver une issue.-- Le montage telle qu'il a été fait en en Charente a été validé par l'administration. Et aujourd'hui on nous dit après un contrôle de la chambre régionale des comptes. Ah bah non, c'est plus possible. Donc vraiment c'est l'amendement. Il a une volonté. Pragmatique, de trouver une solution en tout cas de faire en sorte qu'on.-- Maître dans ce texte. Dans cette loi. Cette problématique pour qu'une solution soit trouvée dans les meilleures conditions. C'est pourquoi moi je j'incite vraiment mes collègues à voter cet amendement.-- Très bien se veut donc mettre aux voix cet amendement avec un double avis défavorable qui est pour.

Il est défendu. Il est défendu l'avis de la commission et sagesse. Voilà et l'avis du gouvernement pareil non défavorables. Oui. Sagesse aussi bien je mais on voit cet amendement qui a un double David ça j'ai skié pour. Qui est contre qui s'abstient il est adopté. Après l'article 37 à monsieur le rapporteur pour le 10 38. De la. Voilà c'est c'est l'amendement qui était annoncé dans le débat sur le PLF qui est d'instituer une conférence de financement des transports publics en Île-de-France avec. La nécessité également de de tenir informer le Parlement des conclusions de cette conférence de financement. Non c'est un avis défavorable. Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir une disposition législative en projet de loi de finances pour prévoir qu'il y a des échanges et des travaux entre l'ensemble des financeurs de des transports publics en Île-de-France. C'est un peu ce qui est prévu là à qui ça demande en plus un rapport au gouvernement. Ce qui est pas très. Normalement. Plébiscité au Sénat et par ailleurs, ça n'est pas le gouvernement qui est responsable des transports en Île-de-France. évidemment. Partant pour participer à des travaux avec la région Île-de-France, ce qu'on est en train de faire, puisqu'il y a des échéances qui arrivent encore cette semaine et je peux vous dire qu'il y a énormément d'échanges en ce moment même entre les différents acteurs de ce dossier. D'accord pour continuer à travailler évidemment avec IDFM avec la région sur des enjeux plus structurant et plus pérenne de financement mais de là à prévoir dans la loi. Qui est une réunion ça ne me semble pas nécessaire donc avis défavorable.-- Je vais donc mettre aux voix après avoir donné la parole à monsieur vol délit. merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Alors c'est vrai qu'il a déjà été présenté à monsieur le rapporteur. Et là ça fait pas le compte Je dis ça au rapporteur général et au ministre.-- La semaine prochaine.-- Il va y avoir des réunions extrêmement importantes qui vont décider que le Pass Navigo en Île-de-France va passer à 90 euros.-- C'est demain. Et on nous dit là il faudrait. Se satisfaire d'une conférence financière. À caractère très urgent avant la fin janvier 2023. Ça c'est la position du rapporteur général donc lui l'augmentation 90 euros du passe Navigo. Et si ça passe demain monsieur le rapporteur général. Les 90 euros et qu'il a pas un mouvement de compensation par l'État à Île-de-France mobilités on ira peut-être au Pass Navigo à 100 euros. Des questions qui sont examinés par l'administration d'Île-de-France mobilités. Donc là on est pris les les usagers des transports parisiens sont pris totalement en otage. Et par ici. Cet amendement qui, on le sait, n'a pas de vertu à apporter une solution dans l'urgence de la situation et par le gouvernement qui arrête pas dire oui, on est prêt à travailler avec la région n'est prêt à travailler car joue les prêtre avec la région. Avec une structure. Qui est en situation d'endettement catastrophique. On l'a dit ici 14 cette année d'endettement de capacité d'endettement mais vous voyez où on est là. On va paralyser les transports de toute l'Île-de-France. Donc ça va avoir des conséquences sur l'ensemble du tissu économique, ça va avoir des conséquences y compris sur le trajet pour aller à la fac ça va avoir des conséquences pour les premiers de cordée dont on a beaucoup parlé ici tous les tâches et les métiers ingrats mais qui font que Paris et

dis, c'est faire du, c'est faire du du du cinéma excusez-moi franchement c'est du cinéma. Vu l'urgence des problèmes des transports. La parole est maintenant à madame Lavarde. Oui juste parce que Monsieur le Ministre, nous a dit, on parle des transports en Île-de-France mais pour dire que les transports en Île-de-France. Aujourd'hui il y a des difficultés qui se posent notamment par les Jeux olympiques et ce que les Jeux olympiques, c'est uniquement une question francilienne. Il y a des questions qui se posent par la mise en place de la Société du Grand Paris est-ce uniquement une question francilienne parce que je rappelle qu'à l'époque où ce projet a été décidé, on l'a qualifiée d'opération d'intérêt national. Alors soit on a changé d'idée sur ce que doit faire ce projet. Mais si ce n'est pas le cas, ça veut dire que la question elle dépasse les frontières de l'de France et le que l'État a un rôle à y jouer aujourd'hui nos transports ont ils ont historiquement été conçu avec un E nodal autour de Paris. Quand on veut aller d'une métropole à une autre, il y a plein de trajet on doit nécessairement passer par Paris. transports de la région capitale. Ils ont aussi un intérêt pour l'ensemble de du périmètre métropolitain. Merci madame la présidente, enfin la situation. Ça Pascal Savoldelli le disait elle est très grave. Elle est. Très difficile et elle va le rester encore pendant des mois pour des millions d'usagers franciliens. Elle représente par ailleurs une vraie menace sur l'attractivité du pays. Tout cela peut coûter aussi en terme de croissance. J'entendais ce matin le ministre de l'économie à la radio qui renvoyait à la question uniquement à la région et à Valérie Pécresse. Valérie Pécresse a interpellé l'État et lui renvoie aussi beaucoup. La balle en réalité vous vous repassez refiler le mistigri entre le gouvernement, la présidente de la région et les républicains. Nous avons voté ici la TVA à 5 5 sur les transports, qu'en restera-t-il dans la suite de la discussion budgétaire. La majorité sénatoriale et le gouvernement ont refusé l'augmentation du versement mobilité que nous proposions suite également à la demande de la présidente de région. Qu'est-ce que cela deviendra dans la suite de la discussion budgétaire. Moi je vois bien comment cet amendement est une. Façon de se dédouaner et de renvoyer les choses à plus tard mais les transports publics en Île-de-France, ils n'ont pas besoin d'une conférence de financement, ils ont besoin de financement et de financement, tout de suite.-- Merci madame la présidente, monsieur le ministre, je partage les remarques qui viennent d'être faites par mes collègues Féroé. Savoldelli, première question, est-ce que la TVA à 5 5 sera maintenu. La situation des transports en Île-de-France est catastrophique. Nous l'avons dit lors du débat, on nous propose aujourd'hui. Cette conférence de financement. Moi je ne suis opposé à aucune conférence de financement. J'ai souvent entendu le rapporteur général nous dire aussi que quand le gouvernement nous renvoyer à des concertations à venir, il y avait un doute, je dois vous dire que j'ai exactement le même doute les solutions, elles sont connues. J'ai défendu dans cette enceinte des propositions formulées par Madame. Pécresse, la TVA à 5 5, elle a été votée. Nous avons défendu une augmentation du versement mobilité. Possible. Elle a été refusée par la majorité sénatoriale et je le dis elle coûtera aussi aux entreprises. Car si le passe Navigo passe à 90 euros. Les entreprises devront en payer 50%. Mais par ailleurs, la désorganisation des transports coûte aux entreprises lorsque les salariés ne peuvent pas arriver à l'heure au travail, donc il y a nécessité d'une solution. Le gouvernement a fait la sourde oreille pendant tous les débats. Il a fait un prêt de milliards et Île-de-France mobilités il pourrait le transformer en dotation. Ça fait partie des demandes. La seule chose certaine, c'est que demander aux citoyens du de dépenser 90 euros pour un Pass Navigo pour être transportés dans des conditions épouvantables et qui se dégrade de jour en jour ça, ça n'est pas acceptable.-- S'il n'y a plus d'explications de vote, je vais mettre aux voix cet amendement du rapporteur de la commission avec un avis défavorable du gouvernement qui est pour.-- Qui s'abstient il est adopté, le 10 14 qui le défend.-- Monsieur de vinasse Monsieur. Féraud. Merci madame la présidente, excusez-moi, je crains pour cet amendement qui était une demande de rapport à l'initiative de notre collègue. Olivier Jacquin, une demande de rapport sur le versement mobilité sur l'ensemble. Du territoire Du territoire national, afin notamment de d'avoir des éléments pour savoir si le versement mobilité pourrait être étendu à des entreprises de moins de 11 salariés et s'il pourrait concerner dans quelle mesure, dans quel objectif. Avec quels moyens les autorités organisatrices de mobilité des espaces peu dense qui sont aujourd'hui dépourvus de base fiscale, je vous remercie. Alors effectivement une demande de de retrait mais je pense qu'on a les moyens. En tous les cas dans le travail des commissions de pouvoir à la fois de travailler sur ce sujet pour une évaluation donc une demande de retrait.

Pour lui, très certainement dire que cet article ne prolonge finalement que. 2 années. Qui plus est sur option la certification par une expertise comptable privé du compte des collectivités concernées. Ce ne sont que 22 collectivités qui ainsi auraient le choix pour nous cela reste inacceptable d'abord le Champ de l'expérimentation remonte à la loi nôtre, cela fait maintenant 8 ans que ce processus est entamé 5 années qu'il a débuté. Seul un rapport d'étape, a été remis, aucun rapport d'évaluation n'a d'ailleurs été rendu. Nous n'avons pas connaissance de dispositions qui entendrait. Cette expérimentation qui nous paraît toujours aujourd'hui dangereuse. 2 régions, six départements, 10 communes 6 EPCI un syndicat. Voilà l'ampleur de cette expérimentation. Je ne peux d'ailleurs m'empêcher de constater que la réduction du nombre de chambres régionales des comptes de 27 à 20. Il faut alors parler de regroupement en langage technocratique se traduit de fait par une baisse de leurs moyens. Les chambres régionales des comptes pouvait s'appuyer sur 1098 effectif en 2009. Elles sont aujourd'hui 10 en métropole, 13 dans les Outre-mer et constate une baisse de 10% des effectifs pour des prérogatives de plus en plus élargie. 1000 agents donc seulement les 2 tiers sont en mesure de contrôler les comptes des collectivités pour au moins 35.000 communes, 101 départements, 18 région 1254 EPCI c'est donc mission impossible. Alors effectivement quand tu la puissance publique est défaillante, faute de moyens. Elle paye ou dans ce qu'a fait payer à des collectivités, des cabinets d'experts comptables privé pour compenser ses propres carences, les missions sont aussi large que l'évaluation de la régularité et la sincérité des états financiers de chaque côté, l'activité la fidélité de sa situation financière et du résultat de ces opérations, une appréciation sur les cycles comptable l'organisation comptable et financière arrêtons donc de transférer des coûts de fonctionnement de l'État vers les collectivités et de fait au cabinet privé.-- Même avis, Monsieur le Ministre, je mets aux voix qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il n'est pas adopté, je me article 37 qui est pour. Qui est contre qui s'abstient il est adopté. Et Monsieur Guerriau, vous êtes, vous avez la parole pour le 11 73

avant le 31 mars 2023. Alors il semble que ce délai est beaucoup trop court par rapport à la date à laquelle la loi de finances pour 2023 sera promulguée. C'est pourquoi nous proposons à travers cet amendement hé bien de prolonger, c'est-à-dire de. De de chèque fixé une date butoir qui soit au 30 juin 2023 et non pas au 31 mars pour éviter ce. Cette contrainte du temps.-- Commission. Favorable, l'avis du Gouvernement. Sagesse je mais on voit cet amendement avis favorable de la commission et sagesse du gouvernement qui est pour.--

Qui compte qui s'abstient adoptée le 11 60. Le président canard à la parole. Oui madame la présidente, monsieur le ministre. Mes chers collègues, nous savons que nous vivons une crise énergétique sans précédent depuis sûrement la seconde guerre mondiale. dans ce cadre, les entreprises publiques locales d'énergie. Font des efforts exceptionnels pour assurer une mission de service public au plan territorial. Elles essayent de contenir la hausse notamment des habitants des territoires desservis. Tant pour les logements individuels que pour les copropriétés que pour les bailleurs sociaux que pour. Les établissements publics, voire même des entreprises. L'objectif étant de faire face à la flambée de l'énergie. Or depuis la fin de l'année dernière, les entreprises publiques locales énergie connaissent. De graves difficultés, comme d'ailleurs les régies de chauffage urbain les rigide d'électricité les où SPL. Les syndicats mixtes et donc l'objectif de cet amendement. Et en fait, de leur permettre. D'ouvrir droit finalement. À ces entreprises publiques locales énergie au PGE résilience. Ah et ainsi de poursuivre et de sécuriser leur demandes de financements en faveur des énergies renouvelables et les technologies sobres et jusqu'à la fin de l'année prochaine donc un message d'espoir pour toutes les entreprises qui aujourd'hui assume une mission de service public exceptionnel et dans un cadre tout à fait. Merci qui. Merci qui. De l'avis de la commission sur cet amendement. Alors c'est, c'est une demande de retrait. J'avoue que. J'ai un peu de mal à comprendre. Le le terme si je le.-- Prends au mot le terme qu'il faut quand même qualifié de. D'entacher la capacité d'endettement je je perçois l'esprit mais je ne pense pas qu'il soit souhaitable d'ailleurs pour aucune entreprise qu'elle soit une entreprise publique locale ou une autre entreprise. D'avoir des dispositifs. Où finalement le PGE et sollicité et si on est en difficulté, on fait en sorte de ne. Pas Pas vraiment tenir compte du PGE. Je crois que c'est ça n'est c'est ne rendre service à personne. Je m'inquiète d'ailleurs de voir ce qui n'était pas possible hier éventuellement devenir possible, j'ai le sentiment que cette échéance de finalement des. De, d'avoir une une franchise de une ou 2 années et puis d'allonger la durée risque. Au regard notamment de la situation que l'on connaît actuellement d'engager. Ou de déboucher sur des désagréments et peut être. Des mauvaises surprises que je ne souhaite pas, je veux dire tout de suite dans, dans quelque temps une donc une demande de retrait. madame la présidente ce le Ministre, mes chers collègues, nous allons soutenir. L'amendement. Dans un article qui est quand même bon on va très vite, on va très vite mais enfin quand même.-- Il y a un encours de 143 milliards d'euros de prêts garantis par l'État. Ah hé bien qu'on aille très vite.-- Et c'est colossal quand même hein.-- Et l'article sur lequel nos collègues nous font l'amendement, il propose de rempiler d'accroître la capacité d'endettement des entreprises via un PGE une nouvelle formule.-- Et cette nouvelle formule est plafonnée à 15% du chiffre d'affaires. Et prévoit un différé d'amortissement de 12 ou 24 mois pour une garantie de l'État.-- Ne pouvant excéder mais ne pouvant excéder 90%. faut faut quand même qu'on comprenne que la première. Réflexion et repose sur les entreprises qui, contrairement aux États ne peuvent pas faire rouler leurs dettes indéfiniment.-- Moi j'attire votre attention là-dessus. Et de report en report est différent différé. Il y a un moment où il faut payer.-- Moi j'attire l'attention hein, on, on va avoir avec ce PGE des bombes à retardement pour une partie des entreprises françaises. Comment ils vont réussir la sortie des prêts garantis par l'État. Donc ça, ça mériterait quand même une réflexion de monsieur le Ministre, pour nous, pour nous éclairer sur comment ces entreprises vont pouvoir se sortir. De s'acquitter de ça et puis la 2ème remarque c'est il y a des absents dans le débat mais, mais je ne dis pas ça pour nous ici, je me permettrai pas.-- Parce qu'ils ont pas lieu de siéger ici c'est des banques privées.-- Elles sont en train de fuir leurs responsabilités quant au financement de l'économie productive et on est en train de se substituer aux banques privées du point de vue leur investissement et de leurs responsabilités vis-à-vis de l'économie productive. Donc à travers cet amendement qu'on va soutenir qui fait preuve de responsabilité. Faut qu'on mesure dans quel, dans quel périmètre, il se tient quoi enfin franchement même en voulant aller très très vite le débat parlementaire. Je rappelle hein. 143 milliards. Oui madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le modeste rapporteur de ces crédits va essayer d'apporter quelques éléments de réponse. C'est que les nouveaux PGE résilience ils sont quasiment pas contracté. Donc on peut faire semblant s'agiter mais la vérité c'est qu'il y a 130 milliards et. Les uns les autres l'ont dit, mais le nouveau puis je résidence c'est 5 milliards et lorsqu'il y aura un des problèmes de défaut, il ne faut pas se mentir et c'est ce que nous avons dit, dans cet hémicycle. Vendredi. Il y a 8 jours. Ce sera pas des problèmes de PGE hein. Ce, ce qu'on est problème d'Urssaf d'abord. Ce sont des problèmes de prix d'énergie d'abord. Alors quand on sera au PGE tout ira bien. Je vous assure. Donc c'est un faux problème, il faut le dire. quand vous parlez aux entreprises. C'est pas ça leur sujet. Leur sujet c'est les prix d'énergie c'est Urssaf qui vont devoir payer et je rappelle que les PGE sont aussi encadré dans un accord européen, donc on ne fait pas tout à fait ce qu'on veut.--

Adopté l'article 37 quater même vote. Adopté l'article 30, quinquet 37, quinquet ce même vote adopté l'article 38 même vote adopté. Et nous passons l'article 39 avec un amendement du président Gontard.-- Merci madame la présidente. étant donné la nécessité d'atteindre un système électrique mondiale décarboné rapidement. L'Agence internationale de l'énergie indique que pour limiter la hausse des températures à 1,5 degrés la production électrique à partir de gaz doit diminuer de 90% d'ici 2040 par rapport au niveau de 2020 et celle à partir de pétrole va disparaître dès 2030 investir aujourd'hui dans ses centrales thermiques dont la durée de vie moyenne et de 30 à 40 ans contrevient donc clairement à ses objectifs. Le gouvernement justifie la poursuite du soutien centrale à fioul et gaz par le fait que celle-ci pourrait améliorer l'intensité carbone du mix énergétique du pays, destination et ce critère sous-entend à tort d'abord que le pétrole et le gaz seraient des énergies plus tolérable d'un point de vue climatique que le charbon et deuxièmement que leur utilisation pourrait être transitoire. Au contraire, nous pensons que soutenir des centrales à gaz ou à fioul aujourd'hui risque de verrouiller le pays dans la consommation de gaz fossile pour plusieurs décennies. Étant donné leur durée de vie 30 à 40 ans, cet amendement vise donc à étant dans l'interdiction des garanties à l'export aux centrales à fioul et à gaz et ça va dans le sens des récentes déclarations du président de la République. Merci.-- Merci.-- Et bien de la commission. Monsieur le Ministre de ma vie je Mezzo cet amendement double avis défavorable qui est pour. Qui est contre ou qui s'abstient. Il n'est pas adopté l'article 39 qui est pour. Qui est contre qui s'abstient adoptée après l'article 39. Monsieur brouillée pour le neuf enfants de suite. Merci. Il s'agit par cet amendement d'accompagner la transformation de notre tissu économique vers un modèle plus durable, plus sobre et plus efficaces conforme à nos objectifs de l'Accord de Paris, il n'y aura pas de transition s'il n'y a pas l'engagement des acteurs économiques aussi sur ce chemin de la transition. Beaucoup s'y engage, cet amendement propose de conditionner le soutien de Bpifrance à la publication d'un bilan carbone et d'un plan de transition pour toute entreprise de plus de 250 salariés. Cette disposition de bon sens pèsera sur le développement des entreprises françaises et les rendra d'ailleurs plus compétitives à l'avenir. Nous proposons pas cette disposition de renforcer également le caractère exemplaire de l'état de décupler la réalisation du bilan carbone pour les entreprises. Mesure qui peine à décoller, malgré son importance cruciale et son caractère obligatoire pour les grandes entreprises.-- Le sénateur Boyer propose de de de de descendre à 250 le seuil de déclenchement de ces dispositifs, bilan carbone plan de transition là où c'est actuellement obligatoire pour les entreprises de 500 salariés et plus. Vous l'avez dit vous-même le dispositif.-- Peine à trouver sa vitesse de croisière donc regardons déjà pour que ce dispositif trouve. Vraiment son bon rythme avant de proposer de descendre à l'échelle inférieure ou de mon point de vue par manque d'expérience et peut-être.-- Par manque d'environnement permettant de travailler sur ces sujets on pourrait ça pourrait entraîner des difficultés d'autant, si vous vouliez. Ce cette question et ses une obligations à des conditions de financement. on utilise souvent le mot transition je pense qu'il faut se donner un temps de période d'adaptation de préparation. Aux entreprises et pour ça il faut évidemment qu'elles aient une perspective et qu'elle soit tu entourées et encadrées. Pour permettre de réussir, donc une demande de retrait.-- m'a dit, Monsieur le Ministre jamais au voir double avis défavorable qui est pour.-- Qui est contre qui s'abstient pas adopté je mon article 40 qui pour. Qui est contre qui s'abstient adopté après l'article 40. Merci madame la présidente. Donc c'est un amendement à l'initiative de notre collègue Nadège avait qui concerne la répartition du produit de la taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer entre différents organismes et cet amendement a pour objectif donc de proposer une nouvelle rédaction ainsi le remplacement des mots à l'exploitation durable des ressources halieutiques part au développement durable de la pêche et des élevages marins permettra d'ouvrir le Champ des possibilités pour les comités tout en répondant aux exigences très encadré réglementairement de la protection des ressources halieutiques et des aides de l'État. C'est une mesure qui est neutre, d'un point de vue budgétaire. Qu'est l'avis de la commission. Qui se propose de d'orienter. Nos une partie de notre activité vers ce que j'appellerais des activités de pêche durable. Je suis enclin à penser que c'est un sujet qu'on peut faire avancer, il faut simplement peut être regarder de quelle manière. Par rapport aux obligations, vous l'avez dit, qui s'impose et notamment aux règles européennes. Comment cette proposition peut se. Situer d'où la demande d'avis du gouvernement. Ses ministres. Oui c'est un avis favorable. Aujourd'hui 35% du produit de la taxe sur les éoliennes en mer est affecté au comité des pêches maritimes et des élevages marins et l'objectif de l'amendement qui est proposée, c'est d'ouvrir les possibilités de financement à d'autres projets, notamment en lien avec les élevages marins ce que la rédaction actuelle du code général des impôts ne permet pas de faire et ça ouvre ses possibilités sans pour autant revoir ou faire évoluer la répartition du produit de cette taxe entre les différents affectataires. Donc c'est un avis favorable.-- Le rapporteur. Avis favorable de, de, de ce fait. Donc je mais on reste un moment double avis favorable qui est pour.-- Qui est contre qui s'abstient. Il est adopté après l'article 40. Un amendement qui monsieur. Merci madame la présidente. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues. Cet amendement s'inscrit au fond dans la continuité du précédent en visant à conditionner les aides publiques accordées aux grandes entreprises à des engagements climatiques contraignants. Je voudrais souligner qu'au moment où les États-Unis engage un immense plan de soutien à leur industrie conditionné à leur accompagnement dans la transition il nous paraîtrait bienvenue qu'en contrepartie des aides versées par l'État et de nombreuses et justifiée en raison de la crise Covid ou de la guerre en Ukraine, les entreprises soient tenus de publier dans les 6 mois qui suivent la réception d'une aide, un bilan carbone renforcées et standardisé couvrant les Scop un, deux sans prise en compte dans le calcul des émissions évitées compenser une stratégie climat articulée autour d'une trajectoire contraignante, un plan d'investissement permettant la mise en oeuvre de cette stratégie. Cette mesure concerne les entreprises soumises à l'obligation de déclaration de performance extra-financière, c'est-à-dire 100 millions d'euros pour le total du bilan 100 millions d'euros également pour le montant Net du chiffre d'affaires et 500 pour le nom de moyen de salariés ces conditions concernent les aides suivantes subventions directes garantie de prêts de l'État. Aides à l'exportation. Crédit d'impôt recherche participation financière par l'intermédiaire de l'Agence des participations de Bpifrance. S'agissant de la participation financière. Nous demandons en outre que celle-ci soit conditionnées à l'attribution, représentant de l'État au sein du conseil d'administration d'un droit d'opposition à tout projet d'investissement incompatible avec les critères de la taxonomie européenne sur les investissements verts.-- Nous avons trois sous-amendements mais ça vol Denis vous les défendez oui. Merci madame Lagarde, la présidente seule mise, mes chers collègues, c'est un sous-amendement là. il y a plusieurs sous sa maman. Nos notre idée le fil directeur, c'est de renforcer les obligations déclaratives des entreprises de plus de 500 salariés en indiquant leur consommation et d'utilisation des produits énergétiques qui nous semble être encore des angles morts dans l'émission dans les bilans d'émission des des entreprises. Voilà, c'est le sens des trois sous-amendements.-- Gain de temps. Mais pas si vous le votez hein parce que bon.-- Quel est l'avis de la commission sur cet amendement, ces trois sous-. Des des sous-amendements pour lesquelles à titre personnel puisqu'ils n'ont pas pu être il été déposée après le passage en commission. C'est certainement un oubli mais je vais rester dans la droite ligne des débats qu'on a déjà eu à plusieurs reprises donc demande de retrait pour les trois sous-amendements comme pour l'amendement.--

Même vote il n'est pas adopté l'article 40 bis. Un amendement du rapporteur. Monsieur le Ministre défavorable je mets aux voix l'amendement de suppression avec avis défavorable qui est pour.--

Oui, j'ai envie dire malheureusement pour notre sujet qui revient chaque année, à savoir celui des relations entre les établissements publics territoriaux et la métropole du Grand Paris, et je dis qui revient chaque année puisqu'en fait. Une loi a été adoptée contre les communes puisque deux fois, avant même que la loi notre la loi MAPTAM soit votée les mères c'était réunion n'assemblée générale et une fois à 94% et la seconde voie à 95%. Il s'était opposé à la métropole du Grand Paris, malheureusement les législateurs n'en n'ont pas tenu compte. Ils ont écrit un texte et puis ensuite il a fallu le mettre en application ce texte prévoyait notamment une montée en compétence de la métropole qui s'accompagner, en parallèle d'une montée en puissance de ses moyens financiers. Sauf que la réalité ne se confortent pas avec la loi puisque on observe qu'en fait le partage des compétences ne s'est pas fait comme l'envisageait le législateur mais que les établissements publics territoriaux ont gardé l'intégralité des compétences parce que bien évidemment quand on parle d'une métropole de 7 millions d'habitants, il y a tout un tas de sujets qui sont beaucoup mieux traités quand ils sont traités au plus près des populations et donc aujourd'hui, on arrive dans une situation où les établissements publics territoriaux. Produisent l'essentiel des services du quotidien quand tu la métropole et c'est d'exister mais vient en doublon de d'autres structures. Dernier exemple que j'ai en tête, elle a créé une structure du tourisme alors même qu'on a déjà un centre un comité régional du tourisme et qu'on a aussi une compétence tourisme au niveau des départements, puisqu'ils sont notamment attributaire d'une partie de la taxe. De ce vient on. Taxe de séjour. Merci. Donc en fait, cet amendement il vient à résoudre un problème qu'on reporte. Chaque année, à savoir celui du transfert de la CFE-qui devait advenir au 1er janvier 2021 qui a été reportée plusieurs fois dans la loi d'ailleurs les sans dire au Conseil constitutionnel, que si la loi est bonne, il faut l'appliquer, si elle est la mauvaise, il faut la corriger donc c'est ce que je vous demande ici c'est de revenir à une situation, chacun sait, soit la CVAE pour la métropole la ACF pour les terroristes. effectivement. Un sujet qui est récurrent.-- Qui paraît pour un certain nombre d'entre nous.-- Compliqué, ça n'est pas un exemple de simplicité. Est-ce que c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le gouvernement. Finalement ne traitent jamais le dossier on on a parlé tout à l'heure des dotations de. Comment dirais-je spécial de de de compensation. S'agissant des métropoles là on voit qu'on a une création sur la métropole du Grand Paris et où finalement les dispositifs permettant de de bien cadrer les financements ne sont. Finalement, jamais mis en oeuvre. Alors il y a une difficulté peut être supplémentaires en tous les cas une question supplémentaire c'est avec la disparition annoncée de la CVAE. Il ne faudrait pas que le gouvernement s'appuie sur ce motif pour dire, écoutez, il faut attendre la disparition pour trouver un dispositif, je crois que ce qui a été évoqué tout à l'heure avec l'arrivée des Jeux olympiques et le rôle et la place de. Paris Région capitale il il est temps de trouver une solution. Monsieur le Ministre, je pense que votre avis est nécessaire. Merci madame la présidente, non mais.-- On le sait tous ici la question du partage des compétences et des ressources entre les communes, les EPT la MGP fait l'objet d'énormément de débats et de discussions depuis 2016. Et je pense que tout le monde partage le fait que l'organisation territoriale existante doit être modifiée. Pour autant, on lui ait pas. Et aujourd'hui il n'y a pas. De schémas cibles sur lequel. Qui aurait emporté une adhésion. Une adhésion assez large et donc c'est vrai que, par conséquent, les lois de finances de 2019 2022, 1021 ont systématiquement. Proroger le schéma trancher tout transitoire de financement de la MGP et des The péter pour sécuriser le financement des acteurs le temps qu'on trouve. Une évolution institutionnelle et qu'il y ait des travaux suffisant pour aller vers une évolution institutionnelle bon on lui ait pas et donc effectivement le texte le PLF pour 2023 qui a été adopté par l'Assemblée. Nationale prévoit dans son article 40 terre de proroger une nouvelle fois de 2 ans. Ce schéma transitoire donc jusqu'en 2024.-- Je le dis, l'objectif c'est donner de la visibilité tout en se donnant la possibilité d'avoir enfin un vrai débat et un vrai travail sur l'évolution institutionnelle moi je me souviens dans le précédent quinquennat il y avait effectivement au début du précédent quinquennat. Une ambition, un souhait du président de la République, du gouvernement d'avancer vers une évolution institutionnelle. Je me souviens que ça avait donné lieu à de nombreuses discussions. Et je me souviens très bien d'en avoir parlé notamment à l'époque avec Patrick Devedjian. Pour le département des Hauts-de-Seine avec d'autres élus. Il y a eu ensuite un certain nombre de dossiers qui sont venus. La réforme des retraites qui n'a absolument rien à voir, mais qui a beaucoup mobilisé le gouvernement la crise sanitaire et ce dossier repasser un peu en dessous de la pile. c'est que dans ce second quinquennat d'Emmanuel Macron. On va avancer sur ce sujet-là et sur enfin une clarification institutionnelle pour la MGP les OPT et plus largement sur la question francilienne. le provoquer entre guillemets en adoptant un amendement qui dès maintenant inscrit dans le marbre une répartition j'en suis pas certain. Mais donc c'est un avis c'est un avis défavorable. En revanche je serais favorable à l'amendement 35 qui est également porté par madame Lavarde et au 1040 de monsieur Husson. Qui est un amendement je pense de, de repli de repli. On va dire. Mais je serais favorable plutôt à cet amendement.-- Monsieur le rapporteur du quel est votre avis. Le siège

qui n'empêche pas de tout changer, je veux dire si on repense le périmètre métropolitain, il faudra tout réécrire parce que si on continue à stratifier du droit sur du droit. On en arrive à ce qui se passe avec l'amendement 35, c'est-à-dire qu'on en oublie même des mécanismes de reversement parce que ce schéma est extrêmement compliqué donc je ne vois pas en quoi dire, on fait la règle du chacun sait soit ce qui permet aussi de venir et répondre à une critique du Conseil constitutionnel puisqu'on vient corriger la loi initiale de 2015 poserait une difficulté. Ça n'empêchera pas dans deux ans, de venir dire qu'effectivement il est nécessaire d'augmenter les moyens de la métropole parce que dans cet intervalle, la métropole a pris de nouvelles compétences. J'avoue que les armes du manque, vous m'avez évoqué pour ne pas retenir cette solution et garder une prorogation de 2 ans je vois absolument aucune différence dans les flux financiers entre les niveaux de collectivités, si ce n'est qu'on ne, on ne tranche pas, on dit juste 2 ans et on on se laisse quand même une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Si le Conseil constitutionnel venait à dire que bon, quatre, cinq années de suite c'est c'est Merci madame la présidente, finalement on a le débat que nous avions tout à l'heure sur la métropole de de de Marseille très clairement le dispositif actuel dysfonctionne. Cependant, je voudrais rappeler quelques éléments qui ont été mis au débat d'abord au sein de la métropole les destins des collectivités sont liées. Deuxièmement cette métropole qui est la plus riche de France c'est une des plus riches d'Europe où la plus riche d'Europe est aussi la plus inégalitaire et paraît par exemple la la CFE-dont on débat aujourd'hui à des taux beaucoup plus élevés dans tous les territoires où la population est la plus pauvre, c'est-à-dire que les entreprises des territoires pauvres payent une CFE plus élevés que les entreprises des territoires plus aisée. je ne fais de procès à personne sur le fait qu'chacun regarde midi à sa porte, mais en tous les cas pour ma part, autant je pense indispensable de voter un statut quoi pour 2 ans parce qu'il n'y a pas de solution, il faut bien que laisser que les territoires puissent continuer à rendent leurs services, autant je pense qu'on ne peut pas prolonger. Et qu'il faut revenir au débat initial de la métropole et donner à la métropole du Grand Paris, une capacité à agir parce que les enjeux climatiques, les enjeux de mobilité. Des enjeux de Gemapi les enjeux de logement ou d'hébergement ne se résolvent pas à l'échelle des territoires et nécessitent des politiques coordonnées. C'est la raison pour laquelle la métropole a été créé. C'est la raison pour laquelle à la Beaujoin d'un effort de simplification et d'un engagement de l'État dans cette réforme. Donc moi aussi j'attends du gouvernement qu'il mette la main à la pâte pour cette clarification, mais pas au détriment de la solidarité donc temporairement maintenant l'existant mais travaillons à renforcer les solidarités et la capacité à agir d'une métropole qui est essentiel sur les sujets climatiques et sur les sujets sociaux. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Sans vouloir allonger les débats mais parce qu'effectivement, même si cela été rapport rappelés par le rapporteur général. C'est un sujet certes complexe mais qui est loin d'être anecdotique pour. Toutes les communes et plus largement pour toutes les populations concernées par cette métropole du Grand Paris, cela a été dit. Également par les intervenants précédents. Depuis, finalement de Minsk 2015 pardon et l'adoption de la loi notre c'est un sujet qui est aujourd'hui récurrent qui n'est toujours pas réglé d'ailleurs vous-même Monsieur le Ministre, vous l'avez reconnu mais à force de renvoyer toujours à l'année suivante. Le problème, en fait on ne le règle jamais nous disons ça d'autant plus tranquillement sur les bancs de notre groupe puisque déjà en son temps, nous n'avions pas voter cette création et nous dénoncions d'ailleurs ce que certains rappellent aujourd'hui. C'est-à-dire que finalement cette métropole du Grand Paris au lieu. De créer des dynamismes Politiques des dynamisme positif qui tireront l'ensemble des communes vers le haut finiront d'accroître les inégalités sociales de la métropole du Grand Paris, en l'état et, et au vu du débat législatif. Tels que les amendements sont cranté. Nous allons bien évidemment voter cet amendement parce qu'il y a un véritable enjeu d'abord à donner de la visibilité pour construire pour investir et pour répondre aux besoins des populations dans les années à venir. Ah flécher le devenir de la CVAE. Pour la la métropole du Grand Paris, la CFE-pour les différents The péter mais enfin bon. Monsieur le Ministre, très sincèrement cette question avoir la prendre à bras le corps. Pas dans un comité technique ministériel, il va falloir la prendre à bras le corps avec les élus de la métropole du Grand Paris et des communes concernées avec la population pour réellement satisfaire de moins demain pardon aux besoins de la population de la métropole du Grand Paris. Monsieur le Ministre. Vous avez dit on n'a pas trouvé mais faut chercher. On n'a pas trouvé la solution mais il faut la chercher effectivement je me souviens parfaitement que le président de la République au début de son premier quinquennat. Eh bien, avait envisagé des choses et puis puis c'est c'est assez perdu dans les limbes mais faut chercher et faut pas chercher à attendent les élections les unes après les autres, en espérant qu'une majorité plus favorable à tel ou tel endroit viennent vous faciliter l'affaire non c'est beaucoup plus complexe que ça. La métropole et il faut s'y mettre et j'ai pas compris qu'elle était vraiment le ministre en charge. De réformer cela et qui vous aviez mis donc quelle est la date monsieur le ministre.-- Alors je vais mettre aux voix, c'est monsieur le rapporteur. Est-ce que vous pourriez nous donner un avis. Voilà. Il vous a pas échappé que après le le la le dépôt d'amendements un certain nombre de nos collègues se sont exprimés, anticipant finalement une forme de sagesse. je crois que c'est important et je voulais simplement dire à notre collègue Daniel Breuiller qu'à ma connaissance. Et selon mes informations et forcément, je les tiens de bonne source. Auparavant, un tiers de la croissance. Bénéficier. Aux EPT. Lorsque. Elle elle elle elle se produisait sur le territoire de la métropole du Grand Paris. Donc c'est aussi pour répondre au sujet des inégalités et je crois que si on veut faire avancer le le dispositif. Monsieur le ministre, il faut un peu poussé les feux. Allô. Et revois cet amendement qui a reçu un avis de sagesse de du rapporteur et un avis défavorable du gouvernement qui pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il est adopté. Et donc les suivants tombe et. L'Arctique et donc maintenant ainsi rédigé, il n'est pas utile de le mettre aux voix et nous passons. Après l'article 40

On est au 692.-- Et qui est identique au Iacovelli qui n'est pas là. Et qui concerne la création de la métropole du Grand Paris.--

d'actualiser la part salaires de TP. Selon le coefficient forfaitaire entre 2015 et la date de révision. Le montant de la dotation de compensation de cette part salaire de TP qui était perçu par les EPCI d'appartenance est aujourd'hui reversé à l'EPT pour les communes concernées dont Alfons dont dont ils font dont elles font pardon excusez-moi, parti à quelques faute d'accord ce soir je m'en excuse. Cet amendement est donc un ajustement technique à la faveur des communes et permet une forme d'équité avec les différents établissements publics territoriaux. Ça va mieux en le disant finalement les villes peuvent bénéficier d'une dépense à la baisse, ce qui n'impacterait pas le budget de l'État ni celui de la mise trop Paul du Grand Paris se présent amendement permet donc de rendre la souplesse aux uns et aux autres dans le montant global des dépenses, nous ne doutons pas que vous nous suivrez.-- un peu. C'est un peu dans le même esprit l'idée en fait et de réintroduire de la souplesse dans les relations entre. Les communes et les EPT notamment dans la partie qui peut être mine minoré ou majoré dans les relations financières entre les deux aujourd'hui. La majoration ou la minoration ne peut excéder que 30%. De des impôts ménages collectés par les communes pour le compte de leur répéter donc le premier amendement le 36, il vise d'une part à actualiser les données qui ont été gelés à 2015 à aujourd'hui, puisqu'on voit bien que les impôts ménages collectés ont cru sur cette, sur cette période, comme la revalorisation forfaitaire des bases. Donc ça c'est l'amendement de repli, le 30 34 il ne fait que ça et le 36 il vient aussi ajouté dans l'enveloppe. La part de la de l'ex-CPS donc la part salaires pour avoir une assiette plus large, donc bien évidemment pour toutes les relations communes péter qui se satisfont du droit existant. Cet assouplissement n'emporte pas de conséquences. Par contre, il existe certains territoires où cette souplesse pourrait permettre d'avoir un soutien plus fort des EPT vers le vers leurs communes notamment certaines qui se trouve aujourd'hui en grande difficulté pour financer leur section de fonctionnement.-- S'agissant donc du fonds de compensation des des charges territorial c'est quand même un flux financiers des villes vers les OPT et se. Présent. Font à des modalités de calcul puisque la fiscalité qui relevait de la TH de l'agglomération ainsi que la compensation salaire cela correspond au montant de base que les villes reverse à l'OPT en gros la MGP reverse à la commune et la commune renverse à l'OPT pour essayer de faire simple. Et lorsque les communes reverse à l'OPT elle verse mais là par rapport à leur valeur de fiscalité de 2015. Et là il y a le problème ça a été soulevée, mais c'est là qu'il a problème, c'est que le PT peu minoré ou majoré de 30% la part du FC c'était sur la valeur 2015 et non par rapport au montant actualisé chaque année en fonction du coefficient forfaitaire d'actualisation donc cet amendement.-- Nous souhaitons que lorsque la commune elle reverse à l'OPT la revalorisation annuelle de la fiscalité selon coefficient forfaitaire entre 2015 et la date de révision soit prise en compte donc c'est aussi une actualisation et ça il y a beaucoup de communes qu'qui demande qu'on reste pas seulement sur le repère de de de 2015. C'est une question d'égalité et d'équité.

Conscient que le le changement proposé ne correspond pas à une actualisation mais en fait. Un changement de fond du mode de calcul du FC FCT dans la mesure où il ne où il semble nécessaire de prochaine refonte plus large du mode de financement des. c'est pas forcément le bon moment, à mon sens, de procéder à cette réforme qui pourrait entraîner des contributions plus élevées pour les communes. Par contre.

Contrairement d'ailleurs à l'amendement 34. Ces amendements supprime aussi la possibilité de faire évoluer à la baisse la contribution des communes et il ne me paraît pas nécessaire de priver les conseils de territoires d'une faculté ou d'une possibilité d'avoir de procéder à un ajustement locale. Et sur les autres c'est également. Non ben c'est bon j'ai fait 80 c'est bon parfait. Merci oui. Même avis défavorable que le rapporteur pour les mêmes raisons sur le 692 le 36 et le 695. Je donne en revanche un avis favorable ou 34 de madame Lavarde qui vient utilement apporter de la souplesse aux mécanismes et aux autres, vous avez été et qui évite de créer des situations de blocage il faudra qu'on ait une réflexion dans le cadre de la navette et du retour du texte à l'Assemblée. Pour voir dans quelle mesure une. Un ajout à l'article si cet amendement est adopté permettrait de garantir et de sécuriser le fait qu'on limite à 5% des recettes réelles de fonctionnement pour la commune. La variation libre du. FC C'est déjà le cas je crois aujourd'hui. Et donc c'est pas présent dans le l'amendement que vous déposez le 34 et donc. Je pense qu'il aura une réflexion d'ici au passage à l'Assemblée. Si cet amendement est adopté pour voir s'il est utile de le préciser ou pas.-- Très bien, madame Lavarde.-- je suis contente déjà qu'a priori un des deux amendements puisse être retenue. Mais le 36 allait quand même plus loin parce qu'on voit bien que la en venant juste actualiser. Les valeurs locatives enfin donc du coup la part, la part des impôts ménages en gros suivant les communes. C'est un peu moins, c'est autour de 50% du du FC c'était ça ne va pas nécessairement pouvoir permettre le transfert de richesses qui pourrait venir des EPT vers les communes en fait il faut bien comprendre que ce dispositif, que ce soit une majoration une minoration c'est un dispositif qui est. Optionnel. Et en fait ça aujourd'hui les les relations entre ville et EPT il y a 12 OPT il a quasiment 12, manière de fonctionner. En fonction des transferts de compétences qui ont eu lieu ou pas à l'intérieur de chacun des EPT et donc on voit bien qu'. Un fonctionnement qui a été prévu de manière très rigide ne permet pas de prendre en compte, par exemple des situations où les EPT ne sont absolument pas intégrer ou quasiment toutes les compétences sont restés dans les mains des villes et ou par contre la richesse économique de la CFE-est arrivé au niveau de l'EPT, donc on a un EPT qui lui a des marges de manière financière à des grosses capacités financières et on a au sein de cet EPT des communes qui elles sont en très grande difficulté à la rigueur elle elles peuvent investir. Mais une fois qu'elles ont investi, elles peuvent plus venir financer leur fonctionnement et donc c'est pour ça qu'on venant élargir l'assiette des reversements de l'EPT vers communes on pourrait leur permettre de pouvoir continuer à investir, donc là on fait un petit petit pas en venant actualiser les valeurs locatives mais c'est dommage en fait de ne pas avoir aussi pris en compte la CPS qui est aussi un peu dans la même veine hein. Aujourd'hui, le problème vient que les EPT non plus de pouvoir de fiscalité. Donc on fait tout transiter par les communes. Mais avant on était quand même sur un schéma qui était quand même plus facile.

Bien je vais donc mettre aux voix ces amendements le 692 double avis défavorable qui est pour.-- Qui est contre qui s'abstient pas adopté le. Est pour. Qui est contre

cet amendement vise à exonérer les communes de moins de 150 habitants du prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources. Le FN GIR le maintien de ce prélèvement met en grave difficulté budgétaire certaines toutes petites communes. Alors que le budget des communes a été fortement amputé depuis 2014. Ces dernières se voient contraints de continuer à contribuer au enfin dire maintenu à son niveau initial souvent la compensation financière devant atténuer la perte de base de la contribution économique CET n'atteint pas le prélèvement au titre du FN GIR et de plus on le sait les charges a augmenté pour tout le monde et à titre d'exemple, je vous cite, la commune de Saint-Mauris, dans la Nièvre, qui compte 68 habitants avec un budget de 58.000 euros et qui versent 7733 euros au titre du FNJ. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Quel est votre avis. Mon avis est une demande de retrait je je ne suis pas certain qu'il faille. Comment dirais-je, exonérer les communes. Quelle que soit leur taille, d'ailleurs. Et et sur le seul critère de la base de population notamment sans faire aucunement référence à un critère de richesse ou à l'évolution des recettes de fiscalité économique. J'ai juste prendre.-- Le cas. Qu'on a évoqué la semaine dernière. De comment dirais-je Ou. Vous l'avez entendu il y a des sommes colossales pour très peu de communes et y compris des petites communes. Voilà donc je pense qu'il faut qu'on soit attentif. Ah c'est possible. Inégalités. Voilà donc c'est pas toujours dans le sens. dirais-je naturel je crois qu'on doit aussi être attentif à ces dispositions donc une demande de retrait.-- Qui contre qui s'abstient n'est pas adopté le 38 madame Lavarde. Oui, alors c'est un problème qui a notamment été évoquée par Philippe mouiller, qui concerne la situation très spécifique des communes qui sont alimentés en énergie par. Un syndicat et aujourd'hui si ce syndicat récupère beaucoup de taxes sur la consommation. La TCF taxe communale sur la consommation finale d'électricité. Il ne peut pas le reverser en section de fonctionnement en commune mais uniquement en section d'investissement et on comprend bien que, aujourd'hui, la situation qui est difficile pour la et pour les communes face à la flambée des prix de l'énergie, c'est devenir payer leurs factures. Donc, l'idée serait que pendant une courte période les syndicats qui ont collecté la. CFE-puisse la reverser en fonctionnement pour que pour que les communes puissent payer leurs factures. c'est une demande de retrait. Je pense que c'est difficile de faire pour une année. Et moi je je comprends et je partage. Les arguments qui ont été défendu je pense que d'abord la finalité de cette taxe elle est aussi. De financer la compétence de l'autorité organisatrice et je, j'ai envie de dire. Faisons confiance peut être à la fois à l'amortisseur électricité et au filet de sécurité en peut être qu'en suivant les propositions sage, raisonnable et de qualité que le Sénat a choisi d'adopter à l'unanimité. On aura pour l'année 2023, les éléments de réponse nécessaire. qui s'abstient. Il n'est pas adopté après l'article 40. Monsieur Cozic. Si madame la présidente. Donc ça. L'amendement proposé par mon collègue Patrice Joly. Qui précise que dans l'exercice de leurs compétences et notamment en ce qui concerne leur politique de gestion de l'espace. Les maires des communes rurales rendent d'indéniables services environnementaux. Or, ces services ne font l'objet d'aucune contrepartie alors même qu'il génère bien souvent des charges pour les communes concernées.-- Il serait opportun de, de réfléchir. La mise en place de paiements pour services rendus pouvant notamment s'inspirer des dispositifs à destination des agriculteurs. Avec le dispositif de paiements pour services environnementaux et donc le le présent amendement propose de solliciter au gouvernement un rapport ayant vocation à proposer des pistes pour mettre en place de tels mécanismes.-- Même avis, Monsieur le Ministre, je mais aux voix qui est pour.-- Qui contre qui s'abstient n'est pas adopté 5 amendements identiques de suppression madame la présidente. Monsieur le Ministre, chers collègues nous avions supprimé lors de l'examen du projet de loi de programmation des finances publiques. Un article assez coercitif à l'égard des grandes collectivités, et on s'aperçoit que subrepticement. Cet article a été réintroduit dans le PLF et donc. Nous proposons la suppression de cet article 40 le le également dans l'amendement de suppression. Je voudrais quand même monsieur nous souvenir que de leur projet de. De programmation des finances publiques pour 2023 2027 et dans la même logique des contrats de corps de 2018 le gouvernement avait alors tenté de faire adopter par le Parlement une seconde génération de contre-Exposition financier entre et collectivités locales. Il était ainsi prévu que celles-ci. À l'effort de redressement des finances publiques, via la l'atteinte d'objectifs de réduction de leurs dépenses réelles de fonctionnement à hauteur de moins 0 5 % par an par rapport à l'inflation prévisionnelle l'état donc c'est aujourd'hui d'imposer aux collectivités locales des efforts auxquels il ne concerne pas lui-même croyant mais pas pratiquant en quelque sorte ce qui est d'autant plus. Contestable que les marges de manoeuvre des élus locaux n'ont cessé depuis d'être réduite au fil des exercices budgétaires. Si les collectivités veulent bien prendre leur part. De l'effort maîtrise. Budgétaire engagée par l'État et de combien y en a moins de rappeler qu'elle dégage un excédent budgétaire et ne pèse donc pas sur les déficits publics ou très peu sur la dette. Leur part dans la dépense publique et d'à peu près 20% et leur poids dans la dette publique globale est de seulement 8,4%.-- Au niveau européen. La dette des collectivités françaises et le poids des dépenses publiques dans les dépenses publiques sont nettement inférieurs à la moyenne européenne. Je rappelle enfin que cette tentative s'était soldée déjà par un échec puisque les parlementaires l'ont finalement rejeté. Le gouvernement tente aujourd'hui avec cet article 42. Quater du projet de loi de réintroduire ce dispositif rejeté. Il porte je l'ai dit porte atteinte au principe de Lyman administration des communes en effet l'encadrement des Budgets de de Cahors va encore plus loin que celui il s'impose donc aux collectivités locales. Et il y a un budget supérieur à 40 millions d'euros.-- Et par conséquent. Pour la même raison je demande le le la suppression de cet article, considérant qu'il n'a pas lieu d'être. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre. À travers effectivement comme d'autres collègues. La suppression de cet article nous pourrions résumer ainsi. Votre message aux collectivités territoriales. Vous n'avez pas aimé les contrats de Cahors, hé bien vous en aurez encore. Je crois que cela vient d'être rappelé vous chercher finalement et c'est peut-être ça l'avantage d'un 49.3 à faire revenir. Par la fenêtre, ce qui a été sortie. Certainement plus dans une, dans une situation bien plus contraignantes. Vous imposer des contrats beaucoup plus de collectivités que précédemment. Et pour autant, celles-ci sont et je ne reviendrai pas ici ce soir dans une situation bien plus dégradée. Moi, je tiens simplement à redire mais très rapidement. Ce que nous avons débattu ici mercredi. Pendant 8h, sur le budget des coliques. La mission collectivités territoriales. Nous devrions fêter en cette fin d'année les 40 ans des lois de décentralisation et finalement à travers cet article. Eh bien vous réintégrer. Un coup de force. Vous avez fait un 49.3 à l'Assemblée nationale et puis vous imposer finalement vous réduisez la capacité à agir des collectivités territoriales cependant et parce que nous sommes un certain nombre à avoir des amendements identiques qui conduiront. Certainement à la comme la même conséquence d'un point de vue législatif tout de même rappeler à la majorité de mes collègues ici et de ceux qui composent la majorité sénatoriale, c'est-à-dire qu'il y a effectivement quelques jours nous avons voté la loi de programmation d'ici 2027. Certes en retirant. Ce type de contrat mais pour autant, quand on accepte l'idée même de pouvoir réduire d'ici à 2027 de 6 milliards les dépenses, hé bien bien évidemment cela permet au gouvernement d'imposer par ce type d'article. Les dépenses auxquelles chacun devrait contribuer et je crois que c'est une toute autre logique que nous devons avoir, c'est-à-dire que quand tu les collectivités territoriales dépenses elles investissent pour nos territoires pour les Françaises et les Français et pour l'avenir de la France. Je ne les ai pas voté dans mon territoire. On nous propose. Des contrats de confiance ou un pacte de confiance pardon le contrat de confiance une. Plutôt ça, ça sentait la publicité. Voilà mais j'ai, on a eu l'occasion de dire également ce ce qu'pensait de ce de ce pacte dit de confiance. Et puis finalement j'ai l'impression, Monsieur le Ministre, pour filer la métaphore sportive que vous tentez là un passage en force. Puisque finalement vous ne. Tenait pas compte même de dans une forme de désobéissance civile de ce que la Première ministre a déclaré au congrès des maires, Porte de Versailles. j'avoue que ça me surprend parce que. Vous savez, trouver dans le PLF. Le Sénat, même quand il est pas bien traité dans le dans l'arrivée d'information avec un amendement qui pesait plusieurs milliards d'euros dans le week-end. Où je pense. On a fait preuve d'esprit de responsabilité et là. Malgré le le flou qui a entouré. Et qui entoure encore un certain nombre de données sur le sujet éminemment sensible et on n'a pas fini de l'énergie et là honnêtement je ne je ne comprends pas, c'est une forme d'entêtement. Je dirais même un peu coupable donc. Je pense que vous allez avoir le même résultat que la première fois lorsque vous l'avez présenté dans le PLF, vous l'avez dit. À mots couverts et notre collègue Cécile Cukierman a repris voilà

Madame brigade et il aller dans le même sens que mes collègues précédemment, puisque cet article ni plus ni moins que la la résurrection des articles 16 et 23 de la loi de programmation des finances publiques dont personne n'a voulu. Il s'agit là d'une d'une atteinte directe. Ça a été dit à la libre administration des collectivités locales par l'encadrement de leurs dépenses de fonctionnement, cet amendement donc propose la suppression de cet article dans la suite logique de ce qui a été votée par notre assemblée lors de la discussion de la loi de programmation aussi. Pouvez-vous, Monsieur le Ministre vous engager cette fois à respecter la volonté du Parlement. Merci. Monsieur le Ministre, quel est votre avis sur. Ces amendements identiques.-- Merci madame la présidente. Moi je vais revenir sur la jeunesse je pas trop long hein, je vous rassure, il est 23h 55. On a eu ce débat d'ailleurs à plusieurs reprises dans le cadre de ce PLF et même dans le. La LPFP mais sur la genèse de ces contrats de confiance. Ces contrats de confiance. Ils sont le fruit. De, j'allais dire dizaines d'heures, mais je crois que c'est le cas de discussion que nous avons eue avec les associations d'élus, avec mes collègues Béchu et Cayeux ces derniers mois pour préparer l'arrivée de la loi de programmation des finances publiques et du projet de loi de finances, avec un premier objectif est un préalable. Tourner la page des contrats de Cahors. Et c'est ce que nous avons fait. Contrairement à ce que j'ai entendu la logique des contrats de confiance n'est pas du tout celle des contrats de Cahors. Et je ne suis pas le 1er à le dire. Puisque l'association des intercommunalités de France elles-mêmes dans un communiqué de presse. A indiqué qu'elle saluait la position du gouvernement, de tourner la page des contrats de Cahors. Je suis d'autant moins le seul à dire que l'association des départements de France, son président François Sauvadet. A publié un. Communiqué de presse indiquant que dès lors que nous retrait. Des dépenses prises en compte dans ses contrats de confiance les AIS, qui ne sont pas pilotable par les départements. Ils étaient favorables à ce dispositif. Et moi j'ai donné tout de suite un avis favorable pour traiter les AIS, de la même manière, j'étais favorable pour qu'on regarde d'autres retraitement par exemple les fonds européens pour les régions peut-être d'autres d'autres dépenses pour d'autres types de collectivités. Donc au contraire, on n'est pas du tout dans la réédition des contrats de Cahors hein parce que il a été travailler avec les associations d'élus ce dispositif. Je ne dis pas qu'elles étaient toutes d'accord évidemment. L'Association des maires de France était opposé, je suis transparent et donc jeudi l'intégralité des positions des uns et des autres, mais en tout cas il est très clair, ça n'est pas la reddition des contrats de Cahors, sinon on aurait réédité les contrats de Cahors, ça n'est pas ce qu'on a fait c'est un dispositif qui part sur la confiance en se disant que on a tous un même objectif, collectivités locales et État c'est de pouvoir continuer à investir dans notre pays. On a besoin que les collectivités puissent continuer à investir, que l'État doit pouvoir continuer à accompagner les collectivités qui investissent et que pour ça il faut qu'on arrive à maîtriser nos dépenses de fonctionnement pour ça qu'on s'est donné un objectif qu'on a voulu donner un objectif dans la loi de programmation. Et pour garantir l'atteinte de cet objectif. C'est là où arrivent les contrats de confiance, on dit on fait confiance aux collectivités locales. Et probablement qu'on aura pas à utiliser ce dispositif. Qui est inscrit dans les contrats de confiance dans le cas où on constaterait que pour une catégorie de collectivités locales il y a. Un décalage très fort par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé. À ce moment-là on ouvre le capot entre guillemets et on regarde s'il y a une ou plusieurs collectivités qui ont tiré leur catégorie ou leur strates vers une dépense importante et on essaie de savoir pourquoi il y a une discussion avec elle et si on se rend compte que il y a pas de raison objective local qui justifieraient alors on s'accorde avec elle sur une forme de retour à la trajectoire. C'est ça les contrats de confiance, ça n'a rien à voir avec les contrats de Cahors. On est allé voir les collectivités je dis on c'est l'État et allez voir les collectivités en leur disant, voilà le contrat voilà ce que vous allez devoir faire vous signez là. Et si vous ne signez pas, c'est l'État qui signe à votre place je je je caricature un peu mais c'est comme ça que ça a été vécu. C'est comme ça que ça a été vécu par les collectivités locales, même si ce n'est pas l'objectif, évidemment, et qui a un gros travail qui avait été fait, on n'est pas du tout là dedans, on n'est pas du tout là dedans et un des enjeux qu'on a pour notre trajectoire financière c'est. De donner de la crédibilité à l'objectif qu'on se fixe. Voilà, et cet outil nous permettrait de donner de la crédibilité à notre objectif. Raison pour laquelle je suis défavorable à sa suppression. C'est vrai que. Il était dans la LPFP la LPFP. A été rejetée à l'Assemblée nationale, elle a été adoptée par le Sénat sans cet article. Je ne sais pas aujourd'hui vous dire si nous aurons une LPFP adopté. Je n'en suis pas certain, pour tout vous dire. Dans ces conditions là. Notre responsabilité c'est d'inscrire dans le projet de loi de finances le plus d'Arctic possible de l'ex- LPFP. Pour nous donner les moyens d'attendre et de tenir notre trajectoire budgétaire. D'ailleurs ça n'est pas le seul article de à la LPFP qui a été repris dans le PLF, l'article sur l'évaluation de la qualité de la dépense publique qui figuraient dans la LPFP. Nous l'avons aussi introduit par amendement dans le PLF parce que c'est notre responsabilité d'introduire le plus de mesures possibles de la LPFP dans le PLF dès lors qu'on pourrait ne pas avoir de LPFP donc avis défavorable sur ces amendements.-- à l'examen du projet de loi de finances, visant notamment la réintroduction dans ce PLF de l'article 23 de la loi de programmation des finances publiques que nous avions supprimé je questionner madame, la Première ministre sur la sincérité du gouvernement dans le débat et son respect du travail du Parlement au moment où nous allons examiner cet article 23 réintroduit sous le titre de 44. Le constat est accablant, vous passez au-dessus des votes, celui de l'Assemblée nationale, celui du Sénat et vous réintroduisez à chaque fois un article qui a été rejetée à la fois par l'Assemblée nationale et par le Sénat le rattachement de ce texte au projet de loi de finances et très contestable, politiquement et même peut être juridiquement enfin c'est plus grave, ça marque une défiance quoi que vous disiez à l'égard des collectivités locales, les collectivités locales n'ont pas besoin de contrat ni de confiance ni de Cahors. Elles ont simplement besoin de confiance, avec ou sans contrat. Elle gère, elle participe à l'investissement public. Vous l'aurez compris, nous voterons bien évidemment la suppression de cet article délétère et ne comprenons pas cette insistance du gouvernement à revenir toujours au-dessus de la parole du Parlement.-- Madame la présidente. Monsieur le Ministre. Quand d'abord félicitations. Ce ministre d'avoir reconnu que le contrat de Cahors était il y a un immense échec un immense four et qu'il ne fallait pas le faire. Bravo et c'est d'ailleurs pour cela que vous nous proposez un nouveau contrat de confiance alors. Le principe de la confiance c'est quand l'Assemblée nationale. Dans sa composition actuelle. Rejette. Légitime. Cette mesure. Lorsque le Sénat. Sa représentativité. Rejettent cette mesure.-- Eh bien la confiance et de respecter le Parlement si vous respectez déjà pas. Le vote du Parlement unanime. Il y a peu de chances que vous respectiez les collectivités locales derrière. C'est pour cela que évidemment nous voulons supprimer en respectant au surplus la parole de madame, la Première ministre. Ce cet article. Oui merci madame la présidente, monsieur le ministre, vous avez évoqué la genèse. Puis après alors je vais vous dire la genèse, hein, vous l'avez déjà expliqué hein. On a changé de ville c'est pas les contrats de Cahors c'est les contrats de Bercy.-- Hé oui hé oui c'est la plus forte baisse de dépenses en volume, du jamais vu. 0,5%.-- Est ce que vous avez omis de dire c'est que c'est vrai qu'une différence, mais après je vais venir aux différents c'est vrai il y a 488 8 villes qui vont être concernées contre 321 avec le contrat de Cahors vous voyez vous nous dites on, on tourne la page, on change tout. Allez, on va jouer au jeu des 7 différences vous en faire cinq pour pas perdre trop de temps. La première, est-ce que dans votre contrat de confiance. Il y a un objectif contraignant des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités.-- Oui est-ce qu'un objectif de réduction de leurs besoins d'auto-financement. Oui et ce qui a une trajectoire de réduction de leur capacité de désendettement. Alors que les collectivités ne représentent que 9% de la dette publique. Oui. Et ce qui est un mécanisme de correction en cas de dépassement de la trajectoire austérité fixé par le préfet.-- Oui. Et ce il y a une reprise financière en cas de non respect de cette trajectoire. Oui et encore oui, donc là franchement si on a rejeté l'article 23 du projet de loi de programmation vous voulez profiter de nous laisser continuer à débattent là alors que, il va y avoir une unanimité et ça a été dit.-- Et là avec le 49 3 en jouant avec telle ou telle appréciation des des des associations d'élus, vous êtes en train de mettre les élus d'ailleurs opposable les uns aux autres, suivant leurs strates de responsabilité, ce qui est pas très responsable du point de vue de l'État et vous allez bafoué l'unanimité du parlement, ça fait quand même un coup double cher à mon avis.-- Monsieur Bonhomme.-- Oui merci au président Wim. Moi je, je comprends que vous essayez d'avoir des propos rassurants. La Première ministre effectivement aux conclusions de du congrès des maires avaient également eu des propos rassurants simplement la la pratique est tout autre et on sait les élus locaux sont d'abord échaudés vous prévalez de l'association de des des intercommunalités. On va pas faire l'exégèse de leurs communiqués de presse en attendant je pense que les 95% des des élus locaux et par leur association sont tout à fait opposé à ce principe de contrat de corps numéro 2 on l'appelle comme veut contrat de Bercy même contrat de Lourdes parce qu'on a parlé de résurrection. On peut, on peut tout évoquer ici. Il n'en est pas, il n'en reste pas moins que ce sont des mécanismes des mécanismes de contrôle quoi que vous en disiez, vous pouvez avoir des propos rassurants et je dois dire ça d'autant plus malvenue que cette année quand même. Si à un moment où on a des difficultés pour construire des budgets, c'est bien cette année Allez voir dans les communes. Comment ça se passe avait tous les éléments exogènes qui leur arrivent tous les jours avec des changements. Réguliers sur l'inflation sur d'autres éléments qui ne maîtrisent pas. Vous avez parlé des AIS pour les départements. Peut-être mais ce n'est pas le cas des communes, c'est pas le cas de de d'autres niveaux de collectivités qui qui vraiment rencontre de graves difficultés donc c'est encore moins. Opportun que les autres années et puis effectivement il y a une question de confiance comme vous, vous étiez le passer par la fenêtre après avoir été. Rejeté par la porte c'est vraiment pas la meilleure façon d'introduire de la confiance dans les relations entre les collectivités et l'État. Oui merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Tout d'abord. Comme l'a fait à mon collègue Savoldelli. Je crois Monsieur mise qu'il faut manier avec prudence. Les éléments donnés. Par telle ou telle association d'élus. Certes, en citant les autres mais on ne le citant pas totalement non plus. Tout d'abord parce que nous savons.-- Malheureusement ou pas. Leur budget ne repose pas sur les mêmes capacités à faire. Parce que leur budget et puisque nous avons cité cité l'association des départements de. France est aujourd'hui. Soumis frappée de plein fouet par un certain nombre de dépenses auxquelles ils sont confrontés pour maintenir les équilibres sociaux dans leur département qui font qu'effectivement il y a des besoins de compensation et qui peut parfois aussi arriver à des formulations d'acceptation mais qui ne veulent pas non plus dire que c'est. Un chèque en blanc à ce qui est fait, je crois. Voilà, nous faisons toutes et tous, ici, de la politique. Donc, faisons très attention à interpréter les uns comme les autres, ceux qui ont dit que tout allait bien et ceux qui ont dit que tout allait mal et l'avantage c'est que comme personne n'a été aussi caricatural dans ses propos que ce que j'aime tenir juste avant. Je crois qu'il faut vraiment écouter avec nuance et modération chaque association d'élus mais sincèrement Monsieur le Ministre. Bien sûr que je ne sais pas les contrats de Cahors. Ça je perds pas de problème. Chacun les appellera comme il veut ici. Mais demain vous allez contraindre et soumettre. Plus de collectivités territoriales pour finalement continuer de faire ruisseler cette idée que la dépense publique serait mauvaise pour l'avenir de notre pays et pour la France. cette la quoi. Nous voterons pour la suppression de l'article 40 quater vous voyez monsieur rapporteur général tout le monde en perdre son latin. Mais à la fin. Les votes seront justes.-- va donc les votes, c'est maintenant. Donc nous allons voter par scrutin public puisque j'ai été saisi d'une demande par le groupe Les Républicains.-- Je rappelle que sur ces amendements. La ville, la commission est favorable et l'avis du gouvernement défavorable. Le scrutin est ouvert.

Le scrutin est clos. Votants 344 exprimés, 340 pour 302 contre 38, le Sénat a adopté.

je sais, on est dans la suite hein, puisque c'est un rapport sur les contentieux administratif. Monsieur le Ministre. Des reprises financière. Et vous rappeler enfin vous rappeler oui enfin on s'en rappelle tous les deux, puisque je vous ai interrogé par exemple sur la situation d'une commune de mon département, la mairie de Villejuif je le seul le ministre. 442.417 de reprise.-- Pour un dépassement de 589.889 c'est la note que le maire de Villejuif dans le Val-de-Marne s'est vu notifier pour un dépassement, écoutez-moi bien.-- Un dépassement de 0 70 %. Vous voyez. il a dépensé 0 70 % des dépenses de fonctionnement de l'année 2019 en plus. Le maire. Est en bas de la douloureuse, excusez-moi de l'appeler comme ça. La signature de l'ancien préfet du département du Val-de-Marne. Ce dernier avait consenti à une ristourne. Il y a eu quand même un geste 90.000 euros après d'innombrables sollicitations toutefois la machine était lancée donc l'étau des contrats de Cahors enserrer les ambitions populaire l'élection d'un nouveau maire de Villejuif.-- Mon collègue Pierre Carzon alors que son prédécesseur avait lui même contractualiser les habitants, les habitants de la commune avait décidé de rompre avec la rigueur et souhaité doter leur ville d'un projet ambitieux et ben ce choix là aurait été enlevé par le contrat de Cahors. On est complètement dans le débat tout à l'heure, le compte administratif servant à la base de la contractualisation a été minoré de près de 400.000 euros. D'autres minoration sont intervenus en 2018 d'aéroport important sur 2019 ont complètement faussé les comptes administratifs en cause dans ce contentieux entre la mairie et l'État. Donc c'était bien un Pack de défiance déjà le contrat de Cahors avant qu'on nous parle du nouveau contrat dit de confiance. Donc il y a peu de procédures contentieuses qui ont fuité dans la presse, Monsieur le Ministre. Donc on voudrait savoir. Où on en est.-- J'ai pu voir une décision du tribunal administratif de Bordeaux qui aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Par exemple le département de la Gironde. Tiens pour aller des départements étaient grâce à la juridiction administrative sûrement un soulagement pour nos collègues. Alors vous demandons interrompu. C'est ce qu'on peut avoir un rapport sur les contentieux entre l'État et les collectivités sur le contrat de Cahors,

Il n'est pas adopté. Après l'article 40 quater un amendement. Merci madame la présidente. Le présent amendement notre collègue Anne Chain Larché propose que le Gouvernement remette un rapport au Parlement sur les modalités de calcul et de recensement de la population dite Insee sur son impact sur les dotations et fonds de péréquation des collectivités locales et sur les pistes de réformes envisageables pour mieux prendre en compte les évolutions de population dans les collectivités locales. En effet la méthode actuelle de recensement de l'Insee qui fournit les données démographiques permettant de déterminer concours financier de l'État envers les communes et défavorable aux communes qui connaissent un accroissement rapide de leur population. Lorsqu'une commune connaît un apport de population importants, les effets ne s'en font ressentir qu'au bout de nombreuses années en ce qui concerne le concours financier de l'État. Or, les communes ont besoin de disposer des moyens suffisants pour pouvoir construire de nouveaux équipements publics et adapter leurs services publics pour le cette population nouvelle sur leur territoire comme des crèches ou des écoles.-- Au moment de la réforme d'ailleurs de la population légale, entrée en vigueur en 2008, il était d'ores et déjà prévu dans la documentation officielle de l'Insee, que bien entendu il sera possible de faire évoluer le système. Dans le temps.-- Par conséquent, et au vu du temps écoulé depuis la dernière réforme, des travaux et études qui ont dû être menées par les services compétents et des impacts majeurs de ces recensements sur le calcul des dotations et fonds de péréquation. Le Parlement doit pouvoir avoir un bilan de la réforme des modalités de recensement et de calcul de la population dite Insee. Aussi, cet amendement propose que le Gouvernement remette un rapport au Parlement sur les modalités de calcul et de recensement de la population dite Insee sur son impact sur les dotations et fonds de péréquation des collectivités locales et sur les pistes de réformes envisageables pour mieux prendre en compte les évolutions de population des collectivités locales. Merci madame la présidente. lorsque vous vous adressez au service de l'Insee puisque cette eux-mêmes qui sont compétents, ils nous expliquent qu'ils ne font que qu'appliquer les dispositions législatives donc et pour éviter une forme de circularité. De l'information mais sans avoir vraiment de solution. Donc je le redis, un avis de sagesse. Si le ministre. Merci madame présidente. C'est un sujet réel et souvent à l'occasion de déplacements je suis interpellé par des maires que je rencontre sur ce sujet. de l'organisation du recensement et de son impact sur le calcul. Des dotations pour la petite histoire encore aujourd'hui où j'étais dans les Pyrénées-Orientales. Un maire m'en a parlé donc je vois bien le sujet. Est-ce que il faut un rapport du gouvernement. Pour répondre à ce sujet.-- Je ne suis pas certain, je pense qu'il faut surtout qu'on arrive à identifier assez rapidement. Des solutions et des propositions pour évoluer. Ça peut passer par un rapport du gouvernement mais surtout il y a aujourd'hui une commission nationale de l'évaluation du recensement là. Qui est présidé par un sénateur. Monsieur Éric Kerrouche. Et qui est explicitement chargée d'évaluer les modalités de collecte des informations recueillies à l'occasion du recensement de la population. Et cette commission présidée par un sénateur a toute latitude pour proposer des modifications aux dispositions législatives et réglementaires relatives au recensement de la population.-- Donc moi, on m'a souvent appris à être défavorables aux demandes de rapport au Sénat, en plus je ne veux pas. Remettre en cause le rôle de cette commission présidée par un sénateur en même temps j'entends le sujet donc j'ai donné un avis de sagesse comme le rapporteur. Mais en tout cas je pense que ce sera important d'embarquer la Commission dans nos travaux.-- Merci madame la présidente, monsieur le ministre. Eh bien écoutez minuit et quart je note j'enregistre et je trouve ça formidable d'avoir deux avis de sagesse sur une demande de rapport. Nous allons bien évidemment voter cet amendement cela d'ailleurs démontre que les jurisprudences parfois. Un peu à marche forcée. La volonté de passer sous certaines fourches caudines un certain nombre d'amendements parce qu'il demande un rapport tombe et s'écroule ici ce soir. Je crois au-delà de la boutade, très sincèrement et je viens d'entendre, y compris, Monsieur le Ministre, les arguments que vous venez d'évoquer. Tout d'abord tous les rapports. Ne sont pas à balayer d'un revers de manche. Avec des avis trop souvent défavorables. Il y a un certain nombre de rapports dont nous avons besoin et on ne peut pas simplement renvoyer comme vous venez de le faire à telle ou telle commission fusse-t-elle. Présidée par par un sénateur, parce que nous nous demeurons convaincus. Que le gouvernement et donc les services de l'État ne sont pas des handicaps. Ne sont pas là pour nous empêcher de faire mais doivent au contraire rempli tout leur rôle de sécurisation de l'action publique et donc quand nous demandons des rapports. C'est justement pour donner à voir pour avoir les éléments et pour permettre au Parlement de faire les choix qu'il faut et pour pouvoir arbitrer en toute objectivité et vous voyez, vous avez balayé très rapidement la proposition d'amendement précédente mais quand on demande à donner à voir là où nous en sommes sur le contentieux par rapport au contrat de Cahors. Ce n'est pas pour embêter ce n'est pas pour pointer tel ou tel problème. C'est pas pour faire plaisir à tel ou tel collègues maires. Avec qui nous serions à proximité. C'est simplement pour donner à voir à un moment donné de l'incohérence de l'incapacité à faire des choix précédents en tout cas, ce rapport va effectivement dans la volonté d'affirmer demain plus d'égalité républicaine dans nos territoires et donc nous le voterons. Qui est contre qui s'abstient. Il est adopté. Je me vois l'article 40 quinquet ce qui est pour. Qui est contre qui s'abstient il est adopté. Nous avons maintenant cet amendements identiques de suppression. Nous commençons par madame Di Folco. Merci madame la présidente. En effet, cet article 40 sexy est-ce qui a été introduit très discrètement par le gouvernement à la faveur du 49.3 vient briser l'accord de financement de l'apprentissage qui a été conclu en octobre 2021. Et qui a été acté dans la loi de finances de 2022 et aussi dans la loi de finances rectificative 2022 et qui a été présenté comme pérennes. Par Madame la Ministre Montchalin alors Ministre de la transformation de la fonction publique et puis même madame Borne, qui était alors ministre du Travail. Le communiqué de presse qui a été rédigé à l'issue de l'accord est très explicite puisqu'il précise, je cite, il s'agit de disposer à compter de 2022, 2 modes de financement pérenne en contrepartie de l'engagement de l'État, les collectivités ont consenti à participer au financement de l'apprentissage par une cotisation supplémentaire de 0,1% de leur masse salariale. 2 82 pour l'année 2022 de 40 millions d'euros, ça représente 50% d'écoute le Cnfpt prenant en charge 10 millions d'euros, l'État 15 millions et France compétences 15 millions, la charge financière qui est prévu pour 2023 est estimé à 90 millions d'euros, compte tenu de l'augmentation conséquente du nombre d'apprentis aussi le désengagement de l'État met en péril le mode de financement, ce qui aura pour conséquence une prise en charge accrue du Cnfpt et des communes alors que les charges qui pèsent sur le budget ne cesse de s'accroître de plus c'est le 2ème. Effet de l'amendement. Il vient supprimer le caractère annuel de la convention d'objectifs et de moyens qui est conclu entre l'État et le Cnfpt plus de débats, plus de négociation possible. Donc cet amendement vise à rétablir les modalités de financement. Franchement monsieur le Ministre rompre uniates unilatéralement un accord n'est pas respectueux et n'est pas acceptable et les collectivités le Cnfpt et les jeunes apprentis mérite plus de considération du gouvernement. Je vous remercie.-- Oui merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, il s'agit d'un amendement identique à celui qui vient d'être défendu excellemment par notre collègue Catherine Di Folco, je rajouterai jusque dans sa grande hypocrisie et non content d'avoir déjà trahi. Sa parole. Le gouvernement n'a bien sûr pas supprimé dans son amendement la cotisation versée par les collectivités qui servait à financer l'apprentissage, donc on a une suppression du dispositif mais on a bien sûr un maintien de la cotisation évidemment. Oui, très rapidement, madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Ça va tout totalement dans, dans le, dans la continuité en en ajoutant. Que le nombre d'apprentis à. A évolué en nombre important. Et. Il y a un sentiment. D'incompréhension de la part des élus qui demandent le respect de cet accord passé été le l'objet de cet amendement. Merci.-- Monsieur de La Et merci madame la présidente. Monsieur le Ministre. Notre collègue di Falco a très bien défendu cet amendement mais moi je voudrais. Rappeler au ministre que si on a parfois quelques contestations sur le soutien à l'apprentissage qui. Qui est parfois un effet d'aubaine et qui ne vise pas forcément la bonne cible. Je pense qu'en matière de collectivités locales, on est dans la bonne cible. On est exactement dans la bonne cible des des jeunes qu'il faut aider et. Moi j'ai toujours plaidé pour ce que qu'on puisse être aidé parce que quand on est maire on a été, vous avez pas encore été maire, Monsieur le Ministre, ça viendra sans doute mais. Je vous le souhaite en tout cas. sachez que quand on est maire on on a envie de pouvoir prendre des apprentis. On est très souvent sollicitée et que là on a un dispositif qui nous aider à le faire, donc c'est vraiment. Pas bien de le retirer.-- Ce seul vol

Ça c'est les mots du président du Centre national de.-- La fonction publique territoriale Cnfpt, François Deluga. En gros, au détour d'un amendement du gouvernement non discuté. Repris par le même gouvernement. Oui, ça c'est le le truc du 49.3 sans vote. Vous décidez de piétiner des mois de négociations avec les collectivités en matière de financement de l'apprentissage. Et là, je vous le dis avec un peu de solennité. Vous nous avez menti.-- Vous nous avez menti le gouvernement. Ce qu'on a voté cet été vous le détricoter l'hiver. OK mais vous nous avez menti madame Borne octobre 2021 cite il s'agit de disposer à compter de 2022, d'un mode de financement pérenne incitatif au recrutement d'apprentis par les collectivités territoriales et soutenable financièrement pour les employeurs territoriaux et des Cnfpt. Imaginez le signal qui a envoyé là et pourquoi nous sommes nombreux ici à demander la suppression de cet article. et je vous le dis c'est c'est c'est irresponsable vis-à-vis de l'échelon local.-- Ça donne une idée de mépris porté aux collectivités et puis un, un faux un faux message sur la question de l'apprentissage, s'il y a bien. Un espace un périmètre où il va y avoir un suivi une attention particulière et une ouverture sur des débouchés, c'est bien par le prisme de l'action des collectivités territoriales, donc franchement il y a là il y a un contrat de confiance à voir avec les collectivités territoriales, sur le rôle qu'elle peut jouer en termes de formation et d'apprentissage.

Alors ce sera une une demande de de sagesse. Monsieur le Ministre. Je, comme j'avais commencé à travailler. La préparation des avis.-- J'avais plutôt compris.-- Qu'il avait une modification dans le financement de des postes d'apprentis dans les collectivités, dont je rappelle quand même que c'est un dispositif qui a une dizaine d'années qui marche plutôt bien, qui doit être à mon avis, encouragés et qui présente un Avantage c'est qu'ils ouvrent sur une palette de métiers et pas forcément. Majoritairement des formation. Type bac plus 5. Je le dis parce que se pose effectivement la question des formations de personnes. Qui n'ont pas toujours. Les qualifications au départ très élevés et donc. Dans l'accord qui avait été trouvé de ce que j'en ai compris alors je ne suis pas allée trouver le bon document.-- D'où la vie de sagesse. Je n'ai pas la certitude absolue mais quand même quasi certaine de ce que le gouvernement s'était engagé. Même et malgré le une cotisation à la charge des collectivités pour participer au financement de l'apprentissage à ce qu'il y ait une part de financement pérenne par l'État et vous l'avez entendu, c'est ce, c'est cet engagement. Que nous demandons. À l'État, qu'ils soient tenu et la moindre des choses c'est de nous assurer que l'État tient aujourd'hui son engagement s'il le fait encore hein puisqu'il est prévu cette année encore, une participation de 15 millions d'euros, à horizon fin 2024 c'est normalement terminée et la manière d'avoir amené un peu en catimini un amendement pour faire disparaître l'engagement dont il n'est plus aujourd'hui pérenne mérite en tous les cas aujourd'hui que vous nous fassiez la lumière et ce sera de mon côté, je leur ai dit, un avis de sagesse.-- Monsieur le Ministre, auquel vous faites référence, oui. Comme quoi, pas besoin d'imprimer. Je l'ai sur mon. Sur mon téléphone pour d'abord moi, je veux dire s'il y a quand même un point sur lequel je pense que l'ensemble des groupes parlementaires dans cet hémicycle, peuvent donner crédit au gouvernement, c'est le soutien à l'apprentissage.-- que six ans maintenant, on a soutenu l'apprentissage comme jamais avec une réforme en 2018 très importante et avec le plan de relance qui a permis de boosté l'apprentissage comme jamais et avec des niveaux attends

dans les collectivités. Territoriales et c'est la raison pour laquelle effectivement a été instituée à la suite d'un accord, un mécanisme de prise en charge par le Cnfpt des coûts de formation des apprentis recrutés par les collectivités locales. Effectivement, le communiqué de presse auquel vous faites référence fait référence à je cite.-- Les collectivités disposeront désormais d'un financement pérenne incitatif au recrutement d'apprentis ce C'est la contribution spéciale à l'apprentissage fixé au maximum à 0 1 % de la masse salariale des collectivités territoriales perçue par le Cnfpt qui est pérenne.-- Quand vous faites référence aux 15 millions d'euros. Je vous invite à remonter un peu plus haut dans le même communiqué de presse que vous évoquez, je cite. L'état prend toute sa part dans ce nouveau système avec un effort financier exceptionnel de 15 millions d'euros cette année. Donc dans le communiqué auquel vous faites référence dans l'accord auquel vous faites référence. Il y a la référence à ces 15 millions d'euros qui sont qualifiées d'exceptionnelles sur une année et en revanche un système pérenne avec la contribution à 0 1 % de la masse salariale qui va de manière pérenne financer l'apprentissage dans les collectivités territoriales. Donc il n'est pas écrit dans ce communiqué, il n'y avait pas été écrit dans cet accord qu'il y aurait chaque année 15 millions d'euros qui viendrait de l'État pour abonder sur l'apprentissage. Ça devait être sur une année en 2022. Qu'est-ce qu'on fait dans le PLF. On le réédite pour 2023. C'était pas prévu au départ c'était pas ce qui était prévu dans l'accord on met 15 millions d'euros en 2023. Dans ce PLF vous ce que vous nous dites c'est il faut, de manière pérenne prévoir maintenant qu'il y a 15 millions d'euros chaque année, il va y avoir une nouvelle convention d'objectifs et de moyens signé notamment entre l'État et le Cnfpt qui va permettre de prévoir peut être de nouveaux dispositifs pour soutenir l'apprentissage dans les collectivités territoriales. Moi je vais pas préempter ces travaux-là et en tout cas. Il n'était pas prévu dans cet accord, que ces 15 millions d'euros soit établie de manière pérenne. Je vous invite à vraiment lire ce communiqué, qui parle de 15 millions d'euros exceptionnel sur une année.-- je vais donc Man, donner la parole à Madame Di Folco ce ensuite un monsieur de La Haye.-- Oui, Monsieur le Ministre, vous parlez de cette fameuse convention vous oubliez de dire et je l'ai moi je l'ai dit dans la défense de l'amendement que cette convention n'est plus annuelle. Ça veut dire que peut-être il y en a. Rue une cette année, enfin l'année prochaine, il n'aura plus après, vous avez supprimé le caractère annuel de cette convention, donc plus de discussion possible. Oui, vous l'avez supprimé, regardez bien votre amendement. Donc ça c'est c'est quand même dommageable, c'est tout à fait dommageable parce qu'effectivement, vous vous engagez encore cette année et on ne sait pas sur les années futures. D'autre part il ne faut pas oublier que ce sont les collectivités territoriales qui ont boosté l'apprentissage bien avant que le gouvernement s'en mêle donc remercions. Enfin, le gouvernement devrait envoyer un signe positif à la jeunesse en disant, on compte sur vos talons et on vous aide à développer vos talents. Oui merci madame la présidente. C'est vrai que moi je n'ai pas le communiqué de presse sous les yeux mais si j'ai bien écouté Monsieur le Ministre, si je l'ai bien compris. Je comprends que ce qui est pérenne dans tout cela, c'est le financement des collectivités locales. Donc ça c'est pérenne. Ça veut dire que vous financez vous en bénéficier. Ça c'est, ça ça peut être pérenne. Par contre le soutien de l'État qui est quand même pas non plus monstrueux 15 millions d'euros, c'est pas par rapport à toutes les sommes que que l'on voit et que, connaît sur le soutien à l'apprentissage qu'il est vrai qu'à qu'a été. À mon avis mal ciblées comme pas mal d'autres dépenses de l'État. Je pense que c'est pas forcément super bien ciblés mais ça alors après, vous nous dites il y a des discussions avec le Cnfpt.

Vous avez dit oui. Les associations d'élus sont favorables à la mise en place d'une cotisation spéciale apprentissage fixé au maximum à 0 1 % de la masse salariale des collectivités territoriales perçue par le Cnfpt.-- Vous avez fait cette citation et puis il y a une omission mais c'est la fatigue. Il y a là et après qu'est-ce qui a marqué. Permettant de financer 50% du coût global de formation mais c'est pas grave que l'évier oublié. C'est pas grave. Parce que qu'est-ce que ça veut dire. C'est que sur 80 millions, il y en a 30 qui vont être payés par l'État et France compétences et il y en a au moins 50 qui vont être payés par les collectivités territoriales.-- C'est pour ça que tout à l'heure avec respect mais de manière responsable, j'ai dit voilà, on nous a menti et quand on nous ment. Bah je peux vous dire que ça c'est assez choquant quoi voilà c'est c'est c'est c'est choquant politiquement et c'est choquant pour le Parlement et c'est choquant pour les collectivités territoriales, parce qu'on leur dit contrat de confiance. Contrat de confiance et puis là on prend une convention, on leur dit l'apprentissage dans les collectivités territoriales mais hop on va vous aider, ça va être pérenne. Ça va vraiment on à vos côtés on à vos côtés a 50 il y a 50% du coût de l'apprentissage qui va être payé par vous.-- Faites le calcul, je ne suis pas sûr que ça soit la même répartition dans les entreprises privées. Très rapidement, il est tard mais je vais quand même répondre à certains points qui ont été qui ont été évoqués. On passe d'une convention annuelle à une convention pluriannuelle.-- S'agit pas dire qu'il y a plus de convention qui est signée avec le Cnfpt. Heureusement, on passe à une convention pluriannuelle, donc au lieu d'avoir une convention caisse chaque année je pense que c'est pas mal en visibilité, surtout quand on parle de ce genre de sujet. Il y aura une convention pour 2023 2024 2025. Qui doit aboutir au début de l'année 2023. Moi, encore une fois je veux pas préempter les discussions qui auront lieu et l'accord qui sera trouvé, je l'espère dans cette convention. En pérennisant une mesure qui n'avait pas vocation à être pérenne. Je le redis et non ça ne voulait pas dire cette phrase que le reste des 50% c'était l'État qui les prenait en charge avec les 15 millions, ce n'était pas du tout ce que ça vaut ce De non laissons sa chance à ces travaux, là on a réédité 15 millions d'euros. C'était pas prévu on avait dit que ce serait que en 2022 c'est prévu en PLF 2023 ce n'est pas dans le texte initial. On l'a ajouté encore une fois, pour montrer qu'on veut donner toute sa chance à cette discussion avec le Cnfpt. Donc je ne vois pas aujourd'hui l'urgence ou l'utilité d'adopter un amendement alors même que les discussions sont en cours.-- Bien ben considérer que la discussion a eu lieu et on va voter. Avis de sagesse de la commission et avis défavorable du gouvernement sur ces cet amendement identiques qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Ils sont adoptés.-- Et l'article et donc supprimer. La l'amendement 114 madame Di Folco. la loi ma trace de novembre 2021 a transféré au Centre de gestion la compétence d'organisation des concours et examens professionnels d'accès au Cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels les catégories A et B en prévoyant que ce transfert s'accompagne du versement d'une compensation financière à la charge de l'État pour un montant équivalent aux dépenses consacrées à la date du transfert par l'État à l'exercice des missions ainsi transférer du code général de la fonction publique prévoit que les cendres de gestion coordonnateur perçoivent la compensation financière relatives à ce transfert et que des conventions sont conclus entre chaque centre de gestion coordonnateur et l'essence de gestion organisateur de ces concours, examens afin de définir les modalités de versement de cette compensation financière. Les conditions de la compensation financière. N'a pu nous n'ont pu être fixé dès la loi de finances 2022. C'est pourquoi le présent amendement a pour objet de fixer ses conditions. Il permet ainsi de diriger la compensation financière uniquement vers les 100 de gestion coordonnateur dans le ressort desquelles sont organisés les concours et examens et en août. Il prévoit la possibilité de résilier réviser le montant de cette compensation financière afin de s'adapter à l'évolution des besoins de recrutement de la filière, de réévaluer de réévaluation ouvrirait la possibilité qu'il ne saurait intervenir avant le 1er janvier 2026 de réviser le montant de la compensation, voire de le diminuer.-- Favorable, quel est l'avis du gouvernement. Pardon défavorable je mais on voit cet, cet amendement 114 avec avis favorable de la commission est défavorable du gouvernement qui est pour.-- Qui est contre. Qui ça. Tiens il est adopté. Donc. On enlève le repli. L'article 40. Qui défend le. MCV.-- Qui est un amendement du groupe défendu. Avis de la commission. Avait du gouvernement. Je mais on voit qui est pour.-- Qui est contre qui s'abstient. Il n'est pas adopté le 482 Monsieur Monsieur Buffet.-- Cet amendement propose de pérenniser la dérogation de à la limite d'âge introduite des dispositions transitoires la 2018 pour une immigration maîtrisée, au bénéfice des médecins contractuels engagés par l'OFI. Je rappelle que cette limite a été fixée à 73 ans et ce jusqu'au 31 décembre 2022, c'est-à-dire dans quelques jours. Or chacun sait que le observe. Toujours de sérieuses difficultés à recruter des, des Lesquels ont été c'était la situation s'aggrave évidemment depuis le Covid et pour toutes les raisons que nous connaissons en matière médicale. Dans ce contexte, il me semble important de pérenniser cette dérogation à la limite d'âge sur le modèle de ce qui est proposé par le gouvernement pour les agents contractuels employés par les pouvoirs publics en qualité de médecin de prévention ou de médecins du travail. J'insiste sur l'importance de la décision et de la mesure à prendre, si on veut que l'OFI au-delà du 31 décembre prochain puisse continuer dans sa mission et singulièrement la mission de santé qui était à sa charge pour les migrants. Monsieur le rapporteur. et il faudrait peut être ne pas trop attendre parce que c'est récurrent depuis plusieurs années, donc il faut au moins se poser la question. Pourquoi sur des métiers comme ceux-là, il y a. À ce point des pénuries récurrentes parce que sinon à un moment donné, on pourrait se trouve en difficulté, on va aussi se dire que. Tant mieux qu'on ait encore des personnes qui acceptent de travailler jusqu'à 73 ans. Mais vous voyez à. À l'heure où on parle d'une retraite qui devrait. Passer au delà de 63 ans entre 63 et 113. Je trouve qu'il y a une marge et ce pas trop à notre honneur. pour rien vous cacher. Dans affiche de banque qui m'a été préparée par mon équipe, il y avait un avis défavorable. Pour envoyer ce débat là au projet de loi sur l'immigration qui va être débattu. Cette mesure et cette dérogation ayant été introduite dans le projet de loi sur l'île dans la loi sur l'immigration en 2018 et en fait, en vous écoutant, en écoutant rapporteur général. J'ai vu que la dérogation s'arrête au 31 décembre 22. Or, je doute que le projet de loi immigration sera adoptée. D'ici là, voilà. Je ne crois pas. Et donc je suis un peu embêtée. Donc je vais en fait j'ai donné un avis de sagesse ce qui nous permettra dans la navette parlementaire et d'ici à l'Assemblée de regarder. S'il y a lieu ou pas de poursuivre cette dérogation.

Pour pousser large des médecins de prévention et de médecins du travail jusqu'à 73 ans.-- Vous savez que depuis 2016 les médecins hospitaliers peuvent rester en activité jusqu'à 72 ans, les agents contractuels employé en qualité de médecin de prévention, par les collectivités. Territoriales peuvent rester en activité jusqu'à 73 ans. C'était le sens de l'amendement là dit défendu de ma collègue Katia pour pourceaux mais parce qu'elle a fait un lien aussi avec un autre. Un autre, une autre loi c'est la loi de finances de la Sécurité sociale pour 2023. Monsieur le Ministre.-- Vous pouvez pas renvoyé seulement à la loi dite sur l'immigration. Vous avez autorisé le maintien en activité des infirmiers et des médecins libéraux jusqu'à 72 ans. Non non non c'est. Vous voyez c'est pas sérieux, on ne peut pas contourner le problème en nous renvoyant une autre loi faut assumer celles que vous que vous avez porté sur la sécurité sociale ou infirmiers et médecins libéraux ont jusqu'à 72 ans, donc voyez on ne peut pas, enfin je vous le dis sincèrement, on ne peut pas annoncer de réforme des retraites qui recule l'âge légal à 65 ans et puis continuer avec ces effets là qui, qui ne vont pas résoudre le problème, moi je veux bien qu'on aille jusqu'à l'épuisement des médecins l'épuisant désir d'infirmer. Voilà et et on n'aura pas la réponse pour couvrir les besoins quoi. C'est le sens de de de la maman qu'on a défendu. Pour Katia pour se présenter pendant le groupe et aussi par Monsieur Buffet. Très bien, jamais aux voit cet amendement. 482. Avis favorable de la commission et sagesse du gouvernement pardon du Qui est contre qui s'abstient il est adopté, je mets aux voix l'article 47 est ce qui est pour qui compte qui s'abstient il est adopté un article additionnel du gouvernement 944. Oui c'est simplement en amont un amendement qui répond à une erreur de codification du Code général de la fonction publique. Merci. Avis de la commission. Qui compte qui s'abstient adopté à partie 47 c'était un amendement. Madame Noël. Oui merci madame la présidente. Il s'agit de deux amendements d'appel de mon collègue Saïd belva. Visant interpeller le gouvernement sur la justice et la rupture d'égalité que représente le fait de n'inclure aucune commune de Haute-Savoie dans la liste des communes ouvrant droit à une indemnité de résidence en effet le code général de la fonction publique prévoit que les fonctionnaires résidant dans une commune où la vie est particulièrement cher dispose d'une prime de résidence d'après une étude circulaire datant de 2001, cette prime est égal à 1 en zone 2 ou 3% zone hein du traitement brut en fonction de la commune de résidence. Cette circulaire fixe également la liste des communes ouvrant droit à cette prime. Cette liste lorsqu'elle a étudié de plus près la en général en zone de des communes où le prix du mètre carré est supérieur de 25% à la moyenne nationale soit supérieure à 3593 euros et en zone hein les communes où le prix du mètre carré est supérieur de 50% à la moyenne nationale soit supérieure à 4300 euros. Cependant, cette liste n'est pas mise à jour de manière automatique et aucun critère n'est clairement posé pour déterminer les communes ouvrant droit à la prime. De ce fait, certaines communes qui répondent aux critères informel ne sont pas incluses dans la liste et n'ouvre donc pas droit à la prime de résidence. C'est particulièrement le cas en Haute-Savoie, dont aucune commune est listé dans la circulaire, alors même que 58% des communes ont un prix du mètre carré supérieur à 3593 euros et parmi lesquels une trentaine ont un prix du mètre carré supérieur à 4300 euros. Cette situation particulièrement injuste et inégalitaire. Pour les fonctionnaires du département qui sont dans une situation identique. Si ce n'est pire que ceux vivant dans les communes incluses dans la circulaire, les parlementaires de Haute-Savoie demande depuis plusieurs années une réactualisation de cette circulaire, alors que la situation ne fait qu'empirer pour le pouvoir d'achat des fonctionnaires qui sont également soumis à une forte attractivité de la Suisse. Je vous remercie.

Accorder d'une façon inégale et les fonctionnaires nommés dans ces territoires subissent des situations de grande précarité. Et. J'd'ailleurs le les préfets de la et de la la Haute-Savoie en 2016, avait indiqué dans un rapport que les difficultés d'accès au logement dans le Genevois français aggrave la situation des services publics au point de les mettre en péril notamment sa continuité dans l'enseignement, la police les le réseau du Trésor public et la santé, le gouvernement s'était engagé devant le Sénat à revoir ce dossier. Considérant que les politiques sociales d'aide à l'accès du logement permettrait à des agents d'avoir accès à un logement adapté pour un coût connu et encadrer notre amendement réitère ainsi la demande de rapport sur la révision du dispositif de l'indemnité de résidence. 25 madame Noël et défendu il est identique, merci. Monsieur le rapporteur. Quel est votre avis sur ces amendements.-- cette ça va être pour les amendements que je qualifie d'appel 162 164 une demande de retrait au profit des 2 autres le 111 et le 165 pour lesquels je rendrai un avis de sagesse. Je pense qu'effectivement il n'est pas normal d'avoir. Comment dirais-je, une situation qui n'a pas bougé depuis 20 ans et puis je, je rappellerai que dans la récente conférence sur les perspectives salariales de la fonction publique. c'est de cette année, en mars 2022, il est dit et même écrit l'indemnité de résidence semble être devenue obsolète, à la fois du fait de son montant trop modeste et de son zonage daté. Monsieur le Ministre, j'invite le gouvernement à remédier assez. Au fait que ces dispositifs date et depuis trop longtemps.-- Oui, avis défavorable sur les quatre amendements que je qualifie les quatres d'amendements d'appel sur ce sujet de l'indemnité de résidence, dont on voit bien qu'elle a effectivement une forme d'obsolescence. Vous savez on est engagé dans un chantier de réforme de l'organisation de la rémunération dans la fonction publique, la réforme de la haute fonction publique a été une première étape, il faut maintenant faire ce travail sur l'ensemble de la fonction publique. La l'indemnité de résidence fait partie de ce qui va être questionné, Il faut rémunérer. Il faut revoir la rémunération de nos fonctionnaires, en tenant compte de beaucoup d'indicateurs et notamment du coût de la vie sur les sur les différents territoires, ça implique de revoir l'organisation de l'indemnité de résidence. Je suis pas certain qu'il faille un rapport du gouvernement spécifique sur ce sujet mais plutôt que le gouvernement en l'occurrence mon collègue Stanislas Guérini qui a en charge l'avenir très régulièrement devant les assemblées pour aborder ce chantier avec vous. Et l'indemnité de résidence en fait partie. C'est pas le seul sujet qu'on va revoir dans cette réforme de la fonction publique.--

Pas adopté. Le 164 même vote.-- Il n'est pas adopté le 111 avis de sagesse de la Commission, avis défavorable du gouvernement ces 2 identique sens de 165. Sagesse de la commission est défavorable du gouvernement qui est pour.

au projet de loi de finances que le gouvernement souhaite supprimer à la faveur du rapport annuel de sur la fonction publique et qui est proposé par la déjà. AFP. Il me semble pourtant nécessaire de conserver cette annexe car les informations contenues dans ce rapport sont beaucoup plus riche et beaucoup plus complète que celle contenue dans le rapport de la DGA AFP qui ne traite pas de toutes les thématiques abordées. Dans le jaune. Il en va ainsi des flux du personnel ou encore de l'apprentissage dans la fonction publique on y revient par conséquent supprimer ce jaune budgétaire priverait le Parlement et l'ensemble des citoyennes une source d'information complète et et d'autre part, la publication des gens budgétaire est prévu par la loi de finances et intervient nécessairement en même temps que le dépôt du projet de loi de finances, si bien que dès la fin du mois de septembre. Le Parlement dispose et l'ensemble des informations nécessaires pour mener son double travail législatif et de contrôle et en revanche, le rapport de la la DG AFP n'a pas de fondement législatif et ça date de publication est très aléatoire et intervient en tout cas trop tard pour permettre le travail parlementaire. De se dérouler dans de bonnes conditions je vous remercie.-- une, une demande de retrait parce que j'ai plutôt dans l'analyse inverse. Avec le rapport de la DGA. AFP. On a des notamment sous forme dématérialisée des données qui a priori sont plus complète que dans le jaune et qui sont la plupart du temps actualisé. De, de manière plus régulière. Donc ce qui m'étonne c'est qu'on ait une lecture différente des documents. merci madame la présidente. C'est un amendement important c'est un amendement transpartisan qui poursuit un objectif très clair, en finir avec l'opacité des prestations de conseil. il est issu. Directement des travaux de la commission d'enquête sur les cabinets conseil de la proposition de loi adoptée à l'unanimité par le Sénat le 18 octobre dernier. C'est aussi un moyen de mettre le gouvernement face à ses responsabilités de lui dire que nous n'accepterons pas qu'il utilise le 49 3 pour dévitaliser notre proposition de loi. L'affaire McKinsey et l'ouverture des enquêtes du parquet national financier des montres que la transparence des cabinets de conseil n'est pas une option, c'est une nécessité. Alors certes le gouvernement a publié un 1er jaune en octobre dernier. Ce document est toutefois très insatisfaisant car il ne Chretien, aucune liste de prestations qui aujourd'hui pourrait me dire quel cabinet de conseil travaille pour l'État pour quelle mission et pour quel montant. La réponse est simple, personne et c'est un problème. Le gouvernement a profité du 49.3 pour créer un jaune dans ce PLF ce dispositif ne nous a pas surpris. C'est le même que celui que le Sénat a rejeté avec force en octobre dernier, le jugeant insuffisant. Alors le gouvernement se cachent derrière le secret des affaires refuse de publier les bons de commande des prestations limitent le périmètre des établissements publics concernés par la transparence en créant un seuil de 60 millions, sorti de nulle part. Tout se passe comme si le gouvernement souhaitait éviter que l'on puisse reconstituer la facture globale des prestations de conseil que la commission d'enquête a évalué à au moins 1 milliard d'euros en 2021. D'aucuns disent, quand c'est flou. C'est pourquoi nous sommes 17 collègues issus de tous les bancs à proposer une véritable transparence sur les cabinets écossais en revenant au texte adopté le 18 octobre dernier ici au Sénat.-- Merci ma présidence une proposition de retrait car satisfait puisque vous le savez, nous avons pris l'initiative de publier un 1er rapport lors du dépôt du projet de loi de finances pour 2023 sans attendre qu'une disposition législative l'impose et ensuite que l'article 40 des de ce projet de loi auquel vous déposer un amendement. Prévoit déjà la création de ce rapport relatif au recours aux prestations de conseil.-- Donc ça me semble satisfait par ailleurs de par la rédaction de votre amendement vous viendriez approuve rire et restreindre les informations qui seraient communiqué. Je ne pense pas que ça soit l'objectif. Mais je vous donne un exemple dans votre amendement et la réécriture que vous faites, vous supprimez la partie 4 cartographie des compétences qui est pourtant présente dans l'article 40 des Siess. Et je précise que cette partie sur la cartographie des compétences, elle faisait partie des recommandations de votre commission d'enquête et nous nous partageons l'objectif. Et donc dans ces conditions là c'est une autre raison pour lesquelles on est défavorable.-- Monsieur le rapporteur. Je vais essayer de vous. Inviter à être favorable, Monsieur le Ministre, parce que moi je remarque que l'amendement vise explicitement outre l'État et si l'établissement public. Les autorités administratives et publiques indépendante la Caisse des dépôts, l'établissement public de santé alors que votre texte se limite aux établissements publics dont les dépenses de fonctionnement sont supérieures à 60 millions d'euros. Donc tant qu'à faire. Autant intégrer le contrôle sur l'ensemble. Oui, monsieur le Ministre, avec tout le respect que je vous dois. Je crois qu'il ne faut pas tourner autour du pot. L'amendement que nous avons déposé avec plusieurs collègues ne fait que reprendre les Arctic III et IV de notre proposition de loi tout simplement et le le jaune que qui nous a été présenté au mois d'octobre. Je suis désolé de le dire mais il y a quand même plein de trous dans la raquette. Donc nous raconte donc avec cet amendement les trous de la raquette et puis si vous voulez, si vous pensez que. Notre amendement est satisfait. Ce que je ne crois pas du tout avec ce que je viens de vous dire, moi je voudrais simplement insister sur un, un fait. Intervenait pour que cette proposition de loi soit le plus rapidement déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale et qu'on on, qu'on ait un débat encore une fois transpartisan et sur le fond. Donc je vous invite à intervenir auprès de vos collègues pour que cette proposition de loi soit déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. Je vais donc mettre aux voix, c'est à mon nom 830 madame Cukierman. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, n'allons pas ravoir ici le débat que nous avions eu à l'occasion de l'examen de cette proposition de loi. je crois qu'il faut être honnête les uns envers les autres. Monsieur le Ministre, vous ne pouvez pas nous dire que l'article telle que rédigée satisfait. Tant aux recommandations de la commission d'enquête qu'au vote qui s'est exprimé ici à l'unanimité à travers la proposition de loi qui en a découlé. Tout d'abord parce que, à travers la rédaction. De cet article. Et donc la création de ce nouveau jaune. Certes qui pérennise dans le temps vous réduisez considérablement. Le périmètre recherché et le périmètre notamment. De publication. Des données. Je reviens pas sur la ligne A excusez-moi 13 qui vise à ne s'en tenir effectivement sur le rapporteur général le disait qu'aux établissements de 60 millions d'euros. Alors que la volonté. D'élargir plus largement. Et puis d'un certain nombre de d'éléments qui ne seront pas contenue dans le jaune. Sauf bonne volonté peut être une année. Mais quel est l'avantage du jaune budgétaire finalement il est d'inscrire et de pérenniser dans le temps pour pouvoir avoir une comparaison d'une année sur l'autre, quelle que soit la bonne volonté ou pas du gouvernement, Vous faites une proposition il y en a une autre, mais en tout cas la proposition que vous faites comme l'a dit la présidente Assassi. Est en deçà. De ce qui a été. Demandé et n'ont pas demandé pour l'exiger mais demander parce qu'au regard de la commission tête d'enquête il y a aujourd'hui effectivement des trous dans la raquette qui laisse passer plusieurs balles et de cela, nous ne voulons plus. Mais donc maintenant mettre aux voix cet amendement qui a reçu un avis favorable de la commission est défavorable du gouvernement qui est pour.-- Qui contre qui s'abstient il est adopté. Je me vois leur dit 42 ce qui pour. Qui est contre qui s'abstient. Il est adopté. L'amendement 945, Monsieur le Ministre.-- Oui, on a adopté à l'Assemblée nationale un amendement qui tire les conséquences de la décrue de l'adhésion de l'Ukraine à la banque de développement, notamment en terme d'augmentation du capital et ici on actualise les montants qui sont prévus pour cela.--

Oui c'est. Vraiment très rapidement c'est pour renforcer le contenu et les modalités de restitution des évaluations de la qualité de la dépense publique. C'est en fait. Tout à fait dans l'esprit en coordination avec la LPFP.--

Il s'agit du bilan des évaluations menées et non des évaluations elles-mêmes et il est nécessaire d'attendre que ces évaluations soient finis afin d'établir ce bilan, qui permet chaque année, identifier des points d'amélioration de ses évaluations. Donc, avis défavorable, parce qu'il ne s'agit pas d'un report à juin des évaluations proposées pour avril dans la LPFP.--

Je vais aux voix avis favorable de la commission défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient est adopté l'article 40. RDC, ce qui est pour. Qui est contre qui s'abstient adopté. Un amendement 11 74 ans monsieur Grand. Et défendu.

Qui est contre qui s'abstient adopté. Le 145. Monsieur Lefebvre.-- Oui madame la présidente, mes chers collègues. Il s'agit par cet amendement de documenter l'impact budgétaire que les retombées en matière économique et culturel tu aurais dû sur la musique enregistrée notamment pour faciliter les échanges sur ce sujet qui pourrait être ne que négocier au niveau européen, ce rapport pourrait notamment évaluer le périmètre du taux réduit l'impact d'une telle mesure sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Les auteurs, les artistes et les producteurs, diffuseurs et les retombées en matière de maintien de la diversité musicale de pouvoir d'achat et d'accès à la culture pour tous et partout sur le territoire. L'avis de la commission. Avis du gouvernement. Même avis je mets aux voix qui est pour.-- Qui est contre Il n'est pas adopté. Article. Amendement 10 44. Monsieur le rapporteur. Suppression de l'article 40 ICS. c'est juste un amendement de suppression de la demande de rapport sur la mise en place d'une TVA circulaire. C'est pas vous surprendre avis du Gouvernement favorable je mais va cet amendement de la commission favorable du gouvernement qui est pour.--

C'est une proposition de retrait puisque la demande est déjà satisfaite. Le code des impositions sur les biens et services, précise que les modalités d'affectation de l'attaque sont prévues à l'article L. 23 33 2 du code général des collectivités territoriales qui mentionne effectivement les EPCI et dans ce cadre. Je pense que l'amendement viendrait alourdir la rédaction de la loi alors même que la demande est satisfaite.------ Qui touche à la compétence donc des agents de des douanes en matière de contrôle de la détaxe de TVA. L'idée. Est. comment dirais-je du rapport que nous avons. Commis. Notamment pour respecter les la protection des données personnelles, on propose que ce soit par un décret en Conseil d'État de préciser les modalités d'application du dispositif qui permet de procéder aux opérations de contrôle. Et notamment pour que ce décret définit la nature des informations consultables, qui l'encadre les modalités de désignation et d'habilitation des agents ayant accès à des informations. Également prévoir. Vous le devinez, les conditions de traçabilité des consultations qui seront effectués réalisé par les agents habilités. Vous savez que dans ce domaine. la protection. À la fois des données des personnes. Et des. Selon les les possibilités offertes aux agents de la douane. Tout doit être parfaitement millimétré bien écrit. Oui, c'est une proposition de retrait. Le code aujourd'hui vers mais déjà la levée du secret fiscal pour l'échange d'informations entre DGFIP et Direction des douanes, vous proposez de d'utiliser l'échange d'informations pour lutter contre la fraude à la détaxe touristique je suis très favorable mais il n'y a pas besoin d'une mesure législative pour cela. En revanche, la création d'un traitement de données supposera un cadre réglementaire est un avis de la CNIL, mais c'est plutôt du réglementaire que du législatif.-- Je mets aux voix cet amendement de la commission avec avis défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il est adopté. Nous avons maintenant le 53 monsieur Oui, cet amendement madame la présidente, poursuit un objectif similaire à celui qui vient d'être évoqué pour l'inscription dans le code général des impôts permettant aux agents des douanes de bloquer les reversements de TVA lorsqu'il y a suspicion de fraude. Il avait de la commission.-- Retrait au profit de l'amendement qu'on vient d'adopter.-- Monsieur le ministre, avis défavorable.-- Ce qu'.-- Vous retirez. Vous maintenez qui est pour.--

Madame la présidente, mes chers collègues. L'atteinte de l'objectif de doublement du nombre d'élèves dans le réseau de l'enseignement français à l'étranger passe nécessairement par des opérations immobilières pour développer les capacités d'accueil des établissements en gestion directe qu'on appelle les C'est pourquoi l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a besoin d'un mécanisme de financement compatible avec les exigences d'un investissement immobilier. Dans la mesure où la EFE reste inscrite sur la liste des organismes divers d'administration centrale les Hodac. L'emprunt lui interdit. Cette difficulté, a déjà été mentionné à la fois dans le rapport sur le contrat d'objectifs et de moyens de la EFE et dans le rapport pour avis sur le programme 185 Diplomatie culturelle et d'influence de la commission des affaires étrangères et de la Défense. Cet amendement néanmoins pour objectif de permettre le développement de projets immobiliers afin de favoriser l'expansion du réseau de l'enseignement français à l'étranger. Le développement d'un projet immobilier peut parfois nécessiter la mise en place d'une entité juridique distincte des établissements scolaires et dédié à celle-ci, l'entité dédiée serait alors lié à l'établissement scolaire. Le dispositif actuel de garantie de l'État ne prévoit pas cette possibilité et cet amant cet amendement entend répondre à ce besoin. Il propose également de ne plus exclure les oeufs GD du dispositif de garantie. Je vous remercie. Oui tout à fait. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet amendement effectivement propose de flexibiliser les possibilités d'obtention de la garantie de l'État pour des entités juridiques.-- De nature privée qui développeraient des étapes des des des projets immobiliers. Pour des établissements homologués mais aussi et c'est une nouveauté pour des établissements en gestion directe, ce qui permettrait effectivement de permettre à l'agence de développer ces établissements ce qui est absolument indispensable et et et et nous comptons vraiment sur. De manière transpartisane sur une adoption de cette proposition qui permet très vraiment un nouveau souffle pour le développement de de notre réseau.-- Alors ces amendements proposent que des structures tierce qui soit d'ailleurs associatives ou privées qui ont signé une convention avec les établissements pour la réalisation d'opérations immobilières puissent bénéficier de la garantie de l'État. Il me semble moi que cet amendement contribuerait à réintroduire un niveau de risque important en permettant à des établissements de créer ou de participer à des structures distinctes de droit étranger qui ne serait donc pas conventionnés avec l'État, sous aucune forme. Et qui pourraient pourtant bénéficier de sa garantie. Par ailleurs, l'amendement propose que ces établissements sous gestion directe, puissent également participer à ce type de montage. Ce qui serait de mon point de vue une spécificité très étonnante. On imagine en effet mal par exemple en France un collège public, créant une entité immobilière privée lever les fonds et obtenir sur ses deniers. La garantie de l'État, sans plus de contrôles. Je rappelle que c'est déjà de la vie que j'avais exprimée lors du PLFR de de 2022. Au cours de l'été le PLFR hein et j'avais un ami un avis défavorable je maintiens cet avis défavorable pour les raisons que je viens d'exposer qui me paraissent. Comment dirais-je exposer justement ces établissements. Elle n'a de gros risques. Monsieur le Ministre, ma vie. Je mais, au revoir.-- Monsieur le comte. serait examiné par la commission qui étudie les possibilités, les les les les demandes de garanties de l'État. Et deuxièmement, je peux vous donner un certain nombre d'établissements qui disposent de moyens éventuellement dans des fondations. Et qui sont bloqués parce qu'ils n'ont pas la possibilité aujourd'hui avec leur statut d'obtenir. Un financement pour leur projet immobilier. Et c'est la seule solution sans risque complémentaires donc je vous demande vraiment monsieur le rapporteur de vouloir bien et tu vouloir étudier avec nous ce ce sujet mais ce qui serait. Le plus favorable, c'est que nous puissions ce soir voter cette disposition et qu'elle puisse être maintenu dans la navette.-- Métro voit double avis défavorable qui est pour.

Ils sont adoptés. qui ont pour objet d'assouplir les conditions d'éligibilité à la prime pour la conversion des véhicules. Ce qu'appelle les rétros fuite les véhicules anciens. Oui un mec qui con convertir véhicules électriques. Dans le 1er cas, il est proposé d'appliquer montant unique de primes par catégorie de véhicules par exemple 5000 euros par véhicule rétro fuité d'second cas, il est proposé d'adopter le montant de la prime à la taille du véhicule. Les véhicules de petite taille se verraient appliquer une prime d'un montant de 5000 euros le véhicule de plus 3 ans, le cinq aurait une prime de 15.000 euros.

madame la présidente. Monsieur le Ministre. L'État s'est engagé à prolonger le dispositif conseiller numérique France service mis en place par la loi de finances pour 2021 et financé dans le cadre du plan de relance via le programme 164. Le projet de loi de finances pour 2023 prévoit une enveloppe de 44 millions d'euros supplémentaires au sein du programme 349 de la mission transformation et fonction publique cet amendement vise à tenir compte de cette évolution des modalités de financement du dispositif qui ne sera plus uniquement abondé par des crédits issus du plan de relance à partir de l'année prochaine, c'est en quelque sorte un amendement de coordination. Il vise par ailleurs à permettre à la elle c'était et la Caisse des dépôts et consignations de signer les conventions avec d'autres organes de l'État souhaitant recourir au dispositif pour accompagner la dématérialisation des services publics.--

L'agence la une. Va entrer en comment dirais-je. Va prendre le dispositif également dans la mise en oeuvre des conventions signées. C'est un rôle qui revenait auparavant à la Caisse des dépôts qui a bien rempli sa mission. Ces 2 dernières années. Pour tout vous dire. Moi j'ai besoin de ce, de l'avis du gouvernement sur cette modification et notamment pour que le gouvernement nous dise. Avec ces changements successifs. Ce qu'il va en advenir des modalités de financement à court et moyen terme de ses conseillers numériques et notamment du rôle de la place ses ventes éventuellement du financement qui le, qui pourrait être demandé ou proposé aux collectivités territoriales.

sur le fait de savoir si on prolongeait ou pas. Cette mesure, si on la pérenniser ou pas. On a fait le choix, l'arbitrage qui a été rendu a été de pérenniser avec une ligne budgétaire doté de 44 millions d'euros qui vont permettre de pérenniser l'emploi de près de 4000 conseillers numérique avec un financement qui est donc désormais dédié et votre amendement. Il prévoit en fait de modifier les conditions de mise en oeuvre des conseillers numériques pour qu'il y ait des conventions conclues entre l'État, la Caisse des dépôts et la haine. C'était moi je n'ai pas d'éléments et dans les questions qui ont pu être posées avant l'examen ou au ministère de la transformation publique m'indiquant qu'il faudrait faire évoluer pour que ce soit plus efficace. Les conditions de fonctionnement. Je pense qu'on a pérennisé le dispositif. Et que donc il va pouvoir continuer à se déployer. Mais il n'y a pas lieu aujourd'hui au sens, enfin de l'avis du gouvernement de faire évoluer le fonctionnement du dispositif qui fonctionne bien. Monsieur le rapporteur de votre avis. Par conséquent.-- Même avis donc jamais aux voix nous l'avis défavorable qui est pour. Monsieur chaises pardon. Oui, mais la présidente, moi je suis ministre. En restant assis en fait vous ne pouvez pas utilisé les crédits les 44 Pillon puisque dans le dispositif. C'est uniquement les crédits du plan de relance qui sont visés. C'est pour ça que cet amendement était fait, c'était pour faire en sorte de.-- Permettre le l'utilisation des nouveaux crédits aujourd'hui vous, vous allez être dans un système qui va être bloqué.-- Je vais donc mettre aux voix qui double avis défavorable qui est pour. Qui est contre Il n'est pas adopté. Le 999, madame Vermeillet. relatives au au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics à modifier les articles L. 401 tiré 5 et L 241 tiré 5 du code des juridictions financières afin de prévoir que la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes puisse dans le cadre de leurs attributions se voir communiquer tout document sans qu'aucun secret protégé par la loi ne puisse leur être opposée. Cette rédaction très large alors que la Cour des comptes et les CRTC dispose d'ores et déjà d'un droit de communication soulève plusieurs inquiétudes quant à la protection des données sensibles et personnelles. Le secret médical, le secret de la défense nationale, elle se crée 5 statistiques en l'absence de tout encadrement le présent amendement prévoit dès lors pour sécuriser cette procédure d'accès aux données et apporter les garanties nécessaires aux personnes potentiellement concernées de renvoyer à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer les modalités d'accès de la Cour des comptes et des CRTC aux documents donnés et traitements couverts par un secret protégé par la loi. Merci. Quel est l'avis du gouvernement. Je mais on voit cet amendement qui a resonné favorable de la commission un avis de sagesse du gouvernement qui est pour.-- Qui est contre qui s'abstient il est adopté. Le 965 Monsieur Salmon. Merci madame la présidente. Cet amendement vise à ce que les services de l'État établissent une évaluation du manque à gagner pour les finances publiques qui résulte de l'utilisation détournée de conventions fiscales internationales conclus avec certains pays et qui sont utilisés pour éviter l'impôt. La fraude fiscale grâce au détournement de ces conventions est estimé à plus de 33 milliards sur 20 ans pour la France et plus de 140 milliards dans le monde. L'amendement et rédigé largement de manière à couvrir également les relations conventionnelles de la France avec les États et territoires non coopératifs afin d'introduire dans les conventions fiscales avec eux les standards les les standards les plus élevés de coopération. De mesures anti-abus et de possibilités de taxation des flux de revenus sortant redevance dividendes intérêts. C'est simplement pour renflouer un peu les caisses de l'État. Merci.-- De monsieur C'est un amendement pour solliciter un rapport sur l'état des conventions fiscales avec le Moyen-Orient. Merci. Quel est l'avis de la commission.-- C'est un avis de sagesse que je qualifierais de sagesse contributive. Sur les deux. Merci. Avis du gouvernement. Oui.-- Avis défavorable, c'est des demandes de rapport il y a eu un rapport sur le sujet en 2015. Ils ne sont pas nécessaire d'avoir un nouveau rapport mais en réalité, je pense que. Indépendamment du rapport, c'est sur la question de ces conventions et du fond que vous voulez interpeller. Le Sénat, je veux dire très rapidement que c'est des conventions qui sont conclues entre États souverains. On ne peut pas les remodeler à notre guise, seul, il faut le faire avec l'autre état. Souverain que nous avons avec 121 convention le second réseau de convention le plus étendu au monde et donc moderniser ses conventions. C'est un immense chantier diplomatique auquel on s'attelle. La la partie. De la problématique consiste à moderniser ses conventions par exemple en révisant les anciennes conventions qui prévoit. C'est l'exemple je crois que vous avez donné un taux nul de retenue à la. Source sur les dividendes. Et je veux dire que c'est moins un sujet manifestement de pays, vous avez cité les États du Golfe qu'un sujet de génération de convention c'est des dispositions des clauses qui a existé dans des anciennes conventions je vous donne un exemple, on est en train de renégocier une convention qui prévoit une clause de ce type avec la Finlande. C'est pas les pays du Golfe. Mais c'est une question de date de convention jusqu'cette convention datent d'une époque où cette clause était quasi systématiquement prévu donc il y a cette renégociation qui en cours sur ces conventions. Par ailleurs, il y a des solutions, notamment dans les accords un ultime multilatéraux comme BEPS pour lutter contre la fraude. En. Et. Pouvant prendre des mesures. Qui viennent s'appliquer sur ces conventions pour lutter contre la fraude. Donc, avis défavorable mais j'espère vous avoir éclairé sur le fond.-- Qui est contre.-- Qui s'abstient. Il est adopté. Me le 52 du coup tombe. Après l'article 40. Monsieur le comte. Le qui a eu le 183. Oui il m'a l'air si madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Depuis 2020 et la pandémie de Covid, le télétravail s'est développée. Il s'est aussi développée chez les travailleurs transfrontaliers.

ne n'aient pas de conséquences en matière de de de de taxation, mais ça n'est plus le cas aujourd'hui. Et, et compte tenu de la difficulté de de de de cette situation mais aussi vous l'avez dit, monsieur le ministre de la difficulté à modifier l'ensemble des conventions fiscales du développement du télétravail. Nous demandons que le gouvernement nous nous remettre un rapport sur la faisabilité. D'une. D'une réflexion. Sur l'application du télétravail chez les transfrontaliers

Avis du gouvernement, ma vie. Je mets aux voix cet amendement avec double avis défavorable qui est pour.-- Qui est contre.--

de fonctionnaires et donc. J'aimerais avoir une réponse un peu plus développé que lors de mon amendement précédent. Il s'agit de fonctionnaires français. Qui vivent à l'étranger. Et qui subissent aujourd'hui. Une interprétation différente. De la part de leur. État de résidence. De la convention fiscale bilatérale entre la France et leur pays de résidence. Je pense en particulier ici lorsque je prends la parole à la Grèce mais surtout à la Belgique. Pour la Grèce une convention fiscale a été renégocié pour en particulier les enseignants du lycée français de Thessalonique de de d'Athènes. Et pour l'ensemble des fonctionnaires qui étaient visés par la nouvelle interprétation par les autorités grecques de la convention fiscale. Il reste encore un certain nombre de cas qui mérite d'être traités et la question aussi de savoir quand est-ce que la nouvelle convention fiscale qui corrige ses problèmes sera ratifié. Concernant la Belgique. Monsieur le ministre, il y a une nouvelle convention fiscale qui a été négocié, qui n'est pas encore ratifié qui ne répond pas aux difficultés des fonctionnaires français, binationaux qui réside en Belgique. Monsieur le ministre, il s'agit de fonctionnaires français.-- Qui sont aujourd'hui doublement taxés parce que la Belgique interprète depuis quelques années la convention fiscale de manière différente suite à. Une décision de la Cour de cassation belge. Alors Monsieur le Ministre, je vous demande et c'est l'objet de ce rapport qu'allez-vous faire pour ces fonctionnaires et nous demandons un rapport sur la manière dont la France réagit à ces nouvelles interprétations des conventions fiscales de certains de de nos partenaires.-- je vais faire. France-, Grèce, France, Belgique. Pour France et Grèce, vous l'avez dit il y a une nouvelle convention qui a été signé en 2022 et par laquelle. Il y a la soumission des revenus des Français résidant grec à une contribution exceptionnelle de solidarité. Qui d'ailleurs ne pouvait pas être assimilé à de l'impôt sur le revenu et qu'il n'était donc pas couvertes par la convention initiale. En ce qui concerne la France et la Belgique et l'imposition des fonctionnaires ayant la double nationalité. Il est clair qu'il a eu un problème de communication entre les 2 pays et malheureusement au détriment de nos fonctionnaires. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a une nouvelle convention convention qui devrait prochainement entrer en vigueur. Vous venez de l'évoquer. Qui doit donc normalement résoudre cette situation et je pense que c'est au gouvernement de nous dire. De manière claire mais pas par le biais d'un rapport l'état actuel des discussions en cours pour répondre, comme vous l'avez sollicité la situation délicate de ces fonctionnaires à la double nationalité. Merci madame présidente très rapidement sur la Grèce. On a signé un nouvel avenant avenant qui rétroactif posiez la question de à partir de quand est-ce qu'il pourra entrer en vigueur. Je vous le précise, c'était important effectivement ce soit d'ici il est rétroactive, donc il s'appliquera sans difficulté sur la Belgique, la nouvelle convention fiscale signée en novembre 2000. 22 lève les incertitudes, elle a été signée. C'est ça lève les incertitudes posées par la convention actuelle en prévoyant clairement le traitement réservé aux rémunérations publiques versées à des binationaux. Par ailleurs, les personnes qui ont fait l'objet des redressements en cause ont été invités à demander l'ouverture de procédure amiable afin de remédier aux situations de double imposition. Donc les 2 conventions nouvellement signés feront d'ailleurs l'objet prochainement de discussion devant le Parlement dans le cadre de leur ratification et donc c'est pour ça que je pense que la rédaction d'un rapport n'apparaît pas opportune vous apporté un certain nombre d'éléments et dans le cadre de la discussion au Parlement sur la ratification. On aura l'occasion de continuer à échanger sur ces sujets.-- Merci madame la présidente. Merci Monsieur le Ministre, pour ces précisions. Je retire donc cette demande de rapport. Et et souhaite Monsieur le Ministre, en en en. En discussion avec vous sur ces sujets parce que de ce que je comprends. Il reste encore des zones d'ombre en particulier sur la manière dont la nouvelle convention fiscale. Négocié entre la France et la Belgique traite l'ensemble des difficultés. Pour l'avenir mais aussi de manière rétroactive, compte tenu des situations difficiles que ces ces personnes rencontrent

nord-africaine enfin africaine de de l'Ouest, suite à la fin du CFA du franc CFA. Un autre rapport qui a trait au régime fiscal des cryptoactifs

Trois amendements pour le 97. C'est une demande de retrait. C'est également une demande de retrait sur le 1148 mais je je pense que le sujet mériterait que le gouvernement nous précise l'état d'avancement des travaux en cours sur le sujet. notamment en souhaitant que le sujet soit abordé au cours du. Prochain budget sachant que je ne suis pas sûr que le, qu'un rapport soit le meilleur moyen d'agir mais qui a un travail qui soient. Voilà. Ça me paraît important. Si le 1148. Alors c'est pas grave c'est le 51 mais c'est le même sujet.--

On passe au 963. Voilà monsieur. Merci le présent amendement propose de mettre en. Place un plan de réduction et de sortie des dépenses ayant un impact néfaste significatif sur le climat ou la biodiversité. La France a pris des engagements parfois insuffisants parfois tardif parfois bienvenu, comme la fin des garanties à l'export, au 1er janvier 2025 tardive comme la fin au 1er janvier 2035 pour les projets gaziers. Il est également essentiel de réduire significativement et de supprimer les niches fiscales néfastes pour le climat. C'est pourquoi, alors que la nouvelle stratégie pour la biodiversité doit être finalisé, nous proposons de concrétiser l'engagement pris de réduire progressivement et de réformer les subventions néfastes à la biodiversité, ce plan devrait identifier les dépenses de l'État les dépenses fiscales et fixé une trajectoire de réduction de sortie Claire et suivi en cohérence avec nos engagements.

L'avis de la commission. Avis du gouvernement. Même avis je mets aux voix qui est pour.-- Qui est contre qui s'abstient et n'est pas adopté. Nous elle le les autres amendements ne sont pas soutenus.-- Monsieur le Ministre. Oui madame la présidente. C'est pour appeler, demander la coordination des articles liminaire et d'équilibre.-- en application de l'article 47 bis alinéa 3 du règlement. Il va donc comme le gouvernement dans ce procédé à une coordination à l'article d'équilibre, à savoir l'article 26 et de l'État a annexe du projet de loi de finances pour 2023

Qui est contre qui s'abstient c'est. Accepter. Et donc nous allons procéder maintenant aux coordination L addition ne peut porter que sur la nouvelle rédaction proposée et on commence donc par votre amendement coordination hein. Monsieur le ministre. Parce Oui donc j'ai présenté à la fois pour l'équilibrer pour le liminaire, si vous voulez bien, comme ça, ça permettra d'aller. Plus vite sur l'article d'équilibre, l'équilibre est amélioré de 29,1 milliards d'euros. Incluant la correction de l'erreur sur la prise en compte du dégrèvement barémique lors de la première partie du PLF pour moins 4,6 milliards d'euros. Vous vous souvenez, dès le lendemain pour la transparence et la clarté des débats j'étais intervenu en reconnaissant qu'il avait eu une erreur. Voilà dans. Le nouvel article d'équilibre. Et il comprend également cet équilibre l'amélioration du solde à l'issue de l'examen de la 2ème partie de 33,7 milliards d'euros je quand même préciser que cette amélioration du solde dans sa 2ème partie est essentiellement due à la suppression de missions entière.-- On peut pas dire qu'il ait 33 milliards d'euros de d'économies qui a été trouvé. Quand on supprime intégralement la mission cohésion des territoires, 17,9 milliards d'euros qui finance notamment les APL ou les maisons France service.-- à la fin ce PLF tels que adopté par le Sénat était le PLF la finale il y aurait plus de financement des APL des maisons France service parce qu'il y aura plus de mission cohésion des territoires. De même sur administration générale et territoriale de l'État, 4, 6 milliards d'euros ça finance le réseau préfectoral mais aussi la confession, la confection des pas des des passeports et des cartes d'identité. On sait que c'est un sujet important pour beaucoup de Français mission agriculture 4 milliards d'euros totalement supprimé Immigration Asile intégration de milliards d'euros pour l'hébergement des réfugiés ukrainiens supprimé et a par ailleurs d'autres économies entre guillemets qui me semble heures. Voilà. pas vraiment structurante notamment de réduire la dotation pour aléas d'un milliard d'euros. Moi je souhaite qu'on ait pas à utiliser qu'on ait le moins d'aléas possible mais je suis pas sûr que ce soit une économie très structurante. Bref, le seul budgétaire suite à ces décisions s'établit désormais à 120 à moins 126,2 milliards d'euros. Et donc je passe sur le liminaire, madame la présidente. En conséquence, le solde du liminaire est amélioré de 1,2 points et s'établirait à 3,7% du PIB. Mais encore une fois je le dis, cette amélioration est factice puisqu'elle est issue de la suppression sèche de plusieurs politiques publiques il y a plus de mystère, l'agriculture et puis le ministère de la cohésion des territoires, donc pas que mais en grande partie, en grande partie, je me suis fait, j'ai demandé à mon équipe de faire le calcul.

De déficit, ce qui n'est pas les quatre si ce que vous aviez prévu dans votre LPFP, je le précise, je le précise. Voilà donc c'était pour la présentation et j'en profite parce que je pense que je ne reprendrai pas la parole pour vous remercier chacune et chacun pour votre participation assidue à l'ensemble des discussions sur ce PLF.-- Merci. Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements.-- Alors je, je propose de rendre la vie à titre personnel puisque ça évite de. Réunir la commission c'est de toute façon ce que ce qui vient d'être présenté tire les conséquences des votes et les conséquences, je dirais comptable et mathématiques. Des amendements de crédit qui ont été adoptées sur le solde budgétaire donc ce sera un avis favorable à titre personnel donc mais que je propose également de suivre. Merci. Je vais donc mettre aussi ça monsieur ça. Ouais. Merci madame la présidence. C'est pour une explication de vote.-- Ça va être très court, voilà. Nos, notre groupe on votera contre. parce que là on est pris dans la mâchoire.-- On avait au départ un projet de loi.-- Qui se qui se positionne sur une baisse des dépenses publiques.-- Alors avec telle ou telle choix et puis on a le Sénat. Enfin le Sénat.-- L'hémicycle. Que je regarde face à moins mais qui est majoritaire, qui a lui. Vous avez eu raison, monsieur le ministre a fait des suppressions de de politique publique.-- Vous voyez, alors la question de du calcul lui-même nous avons il est raisonnable, il est sincère, il y a aucun problème mais c'est pas un problème de calcul, c'est un problème de fond de fonds de comment on approche la question des politiques publiques, celle de l'État mais aussi des politiques publiques, des collectivités territoriales qui encore ce soir encore ce soir ont été peu respectées. Voilà donc on votera contre.-- S'il n'y a pas d'autre explication de vote je mettre aux voix d'abord l'amendement de coordination. Inquiet pour.

l'examen des articles de la seconde partie du projet de finances pour 2023. La prochaine séance aura lieu à mardi, mardi 6 décembre à 14h 30 pour les explications de vote sur l'ensemble du projet de loi de finances et le scrutin public. À la tribune. Je vous remercie. Et bien sûr. Et la séance est levée.